La séance est reprise en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques, a émis lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable 18 voix pour, 2 contre à la reconduction de Monsieur François Jacq, aux fonctions d'Administrateur Général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture visant à combattre le harcèlement scolaire. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Thomas dessus pour le groupe écologiste solidarité territoire pour 4 minutes.

ils font face au moins une fois dans leur scolarité, le harcèlement scolaire est un fléau pour notre pays, des cours d'école aux réseaux sociaux jusque dans les jeux vidéo, les victimes n'ont aucun répit, avec parfois des conséquences terribles et définitive ce drame nous oblige et nous devons leur apporter une réponse, c'est l'objet de cette proposition de loi. Fruit des travaux d'Erwan Balanant à l'Assemblée nationale, ce texte fait le choix, tout d'abord de la reconnaissance d'un nouveau droit d'un principe essentiel: celui d'une scolarité sans harcèlement. Pour faire respecter ce droit, il a créé un nouveau délit : celui de harcèlement scolaire a ressorti d'un panel de sanctions très élevé entre 3 et 10 ans d'emprisonnement et 45 à 150000 euros d'amende selon la gravité, c'est sur ce point particulier que porte en grande partie les désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat notre haute assemblée a fait le choix de ne pas créer de délit spécifique, mais d'intégrer le harcèlement scolaire comme circonstance aggravante du harcèlement moral, nous avions soutenu en première lecture cette réécriture et nous n'avons pas changé de ligne, nous considérions le quantum de peine du délit de harcèlement de l'Assemblée nationale, beaucoup trop élevé pour les mineurs, surtout lorsque le harcèlement est un phénomène de groupe se serait quasiment inapplicable, nous comprenons l'ambition de l'Assemblée nationale de vouloir avec ce nouveau délit permettent une meilleure caractérisation des spécificités de ces agressions par les forces de l'ordre et d'attirer encore davantage l'attention de la société des élèves et de la communauté éducative sur le sujet, mais nous estimons que l'enjeu réside plutôt dans la formation de tous les acteurs concernés dans l'identification, la détection et la prévention, et je l'ai dit, en première lecture et certains l'ont dit avant moi, l'état de délabrement de la médecine scolaire dans notre pays est un frein à ce processus, les médecins, infirmiers et infirmières scolaires pourraient être les vigies qui nous manque tant, avec un peu moins de 1000 médecins scolaires et de 7500 infirmiers, infirmières scolaires pour 12,5 millions d'élèves dans notre pays soit un médecin pour 14000 élèves et un infirmier ou infirmière pour 1600 élèves cette tâche est tout simplement impossible d'autres désaccords entre les 2 chambres, on a aussi vu le jour, notamment sur la reconnaissance claire du cyber harcèlement dont l'Assemblée nationale ne veut pas ou encore les informations du tissu associatif, l'implication des Cruz ou les stage de responsabilisation, à la vie scolaire, ont cette fois-ci, le Sénat ne veut pas, mais c'est la suppression du délit de harcèlement qui a soulevé le plus d'incompréhension, surtout chez certaines associations de victimes, il aurait été plus sain et salutaire d'en débattre à nouveau lors de cette deuxième lecture, mais notre rapporteur à déposer une question préalable sur ce texte, nous le déplorons refuser le débat n'est jamais une solution surtout des sur des sujets aussi graves et sensibles où nous aurions souhaité discuter ce texte confronter les visions des 2 chambres pour lever les ambiguïtés et incompréhension, nous aurions pu voter le texte imparfait, et trop répressive de l'Assemblée nationale mais c'est pourquoi nous voterons contre cette motion préalable, je vous remercie.

minutes. Ce président, Monsieur le Ministre, c'est le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Républicains est évidemment favorable à toutes les mesures visant à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire qui demeure trop souvent silencieux, et dont les conséquences sont destructrices, conscient de ce sujet préoccupant, le Sénat avait d'ailleurs diligenté une mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement c'est fort de ce travail que nous avons adopté plusieurs mesures concrètes et opérationnelles dans l'examen du texte, mais force est de constater que l'Assemblée nationale en refusant d'y accéder, s'est contenté de conférer au texte une valeur symbolique. Comme vous le savez, la commission mixte a échoué sur un point d'achoppement pour nous majeur : la création de délit spécifique de harcèlement scolaire qui viserait aussi bien les élèves que les adultes travaillant au sein de l'établissement, or nous estimons qu'il n'y a pas lieu de viser des adultes comme de potentiels, auteur de cette infraction, point sur lequel d'ailleurs, Monsieur le Ministre, le gouvernement s'était également déclaré défavorable lors des discussions sur la loi, école de la confiance d'une part parce qu'il nous semble évident que d'éventuelles menaces ou abus d'un adulte, ce rendez-vous ne relève pas du même type de situation que le harcèlement qui peut exister entre élèves et ses éventuelles actes de malveillance provenant de personnels adultes au sein de l'établissement scolaire sont d'ores et déjà réprimés pénalement ou sanctionné sur le plan administratif et disciplinaire, d'autre part parce que, avec cette disposition, nous pouvons nous interroger sur le sens du message envoyé aux enseignants, à un moment où leur autorité souvent remise en question, tant par des élèves que par des parents, en effet, nous ne constatons les parents sont de plus en plus prompt à intervenir dans le quotidien scolaire des enfants, alors à partir de combien de mauvaises notes ou de punition pour devoir non fait certains parents, vos qu'il appelait au harcèlement si mes chers collègues, je crains fort que la nouvelle définition ouvre la porte à toutes les dérives et envoie aux équipes pédagogiques, un bien mauvais signal finalement la création d'indécis spécifique de harcèlement scolaire et la disposition centrale du texte sur ce point, nous rencontrons un nouveau désaccord en effet la loi consacrant déjà le droit à une scolarité sort c'est et disposant de l'arsenal juridique nécessaire, pourquoi une telle surenchère au-delà de sa valeur symbolique, ce texte semble surtout avoir une valeur politique régis par l'approche d'échéances électorales importantes dans ces conditions, parvenir à un texte commun semblait bien difficile si le maintien de l'enfant dans son milieu scolaire et par principe, la voie privilégiée, il peut être nécessaire, voire indispensable, au regard de son état psychologique de l'éloigner au plus vite, ainsi j'avais personnellement proposé de mettre rapidement à l'abri, un enfant en danger en permettant aux parents le recours en cours d'année à l'instruction, en famille ou à l'enseignement à distance, dans le même esprit, nous avions élargi les conditions d'une déscolarisation d'urgence en cas de plaintes déposées et nous avons fixé la nécessaire prise en considération de la parole de l'enfant, hélas, ces dispositions ont été supprimés en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'examen du texte par le Sénat aura néanmoins permis plusieurs avancées : le dépistage du harcèlement par les visites médicales obligatoires ou la reconnaissance de l'importance du travail des assistants d'éducation, vers le cyber harcèlement, hélas, partie intégrante de la vie des élèves, il est regrettable que les députés et supprimé la plupart de nos apports, vous l'avez compris, nous ne sommes pas satisfaits de ce texte dont les avancées restent trop limités, nous ne pouvons acter et regretté la disparition des améliorations que nous avions apporté et notre désaccord sur 2 points fondamentaux : la mise en cause des enseignants et la création de délit spécifique qui explique que nous soutiendrons la motion tentant à opposer la question préalable, je suis par ailleurs convaincue que l'efficacité de la lutte contre le harcèlement scolaire repose au moins sur une intervention législative que sur des mesures de terreur et des moyens pour les mettre en oeuvre, que dire du manque criant de médecins scolaires, d'infirmières, de psychologues, pourtant les plus à même de repérer la détresse de l'enfant, ce sujet est pour moi essentiel : il est la première réponse que le gouvernement aurait dû apporter en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement c'est donc avec un sentiment d'inachevé malgré la qualité du travail de Jacqueline Eustache-Brinio et d'Olivier Paccaud, que nous suivrons-nous rapporteur en concluant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue. La discussion générale est Close, nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable et pour défendre cette motion, la parole est à monsieur Olivier Paccaud pour 10 minutes. monsieur le président, Monsieur le Ministre, très chers collègues. Nous souhaitons tous, tous, une lutte renforcée contre le harcèlement scolaire intégrant toutes ces dimensions avec des mesures efficaces compréhensible donc acceptable par les élèves. C'est pourquoi la Commission a fait le choix de déposer cette motion. En effet, nous estimons que ce texte rate sa cible. Article 1er, l'Assemblée nationale a fait le choix de rétablir sa définition du harcèlement scolaire incluant les faits commis par un adulte sur un élève. De manière constante. Le Sénat s'est opposée à cette extension du périmètre du harcèlement scolaire est-ce dire que nous sommes contre une sanction de tels agissements par un adulte, évidemment non, mais le droit actuel permet déjà de sanctionner administrativement et pénalement un adulte comme étant de tels actes, en revanche, dans le contexte actuel de défiance de la société envers l'institution scolaire, comme vient de le dire, Max Brisson, cette extension du périmètre participe à l'affaiblissement de l'école aujourd'hui, un enseignant sur quatre Monsieur le Ministre, se demande s'il n'aurait pas mieux fait de choisir une autre voie professionnelle que l'enseignement. Alors que les enseignants se plaignent régulièrement d'un manque de soutien de leur hiérarchie, ce pas de vague que votre ministère du combattre. Mais bon, ils ont du mal à voir les traductions au quotidien, quel message va envoyer cette nouvelle définition du harcèlement scolaire. Celui d'une suspicion généralisée sur les personnels de l'Éducation nationale je regrette vivement le revirement de position du gouvernement sur le sujet, monsieur le Ministre, vous déclariez ici même il y a moins de 2 ans, à l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, je vais vous citer, il est bon de distinguer les faits qui relèvent de l'action d'élèves envers d'autres élèves, autrement dit de mineurs envers des mineurs de ce qui relève de l'action d'adultes vis-à-vis de mineurs, c'est un problème distinctes qui ne s'apparente pas forcément au harcèlement, nous n'avons pas intérêt à mettre ses actions répréhensibles sur le même plan, vous parliez d'or il y a 15 jours, lors de la première lecture de ce texte, c'est la position de Madame Moreno qui vous représentait était tout autre, je la cite. L'enjeu de cette proposition de loi et de protéger les enfants contre le harcèlement, quel qu'il soit, quelle que soit la personne ayant commis les faits de harcèlement, qu'il s'agisse d'un autre élève ou d'un professionnel qui travaillerait au sein de l'établissement. Comment expliquer ce virage à 180 degrés jouera-t-il une forte hausse en 2 ans du nombre d'adultes travaillant dans un établissement scolaire est soupçonné de participer à des phénomènes de harcèlement. Les auditions que j'ai pu mener dans le cas de cette proposition de loi disent tout et le contraire. En revanche, cette nouvelle définition participe à l'affaiblissement de l'autorité du professeur. Une boîte de Pandore s'ouvrent. J'en viens maintenant au 2ème, point de divergence majeure avec l'Assemblée nationale la création d'un délit spécifique prévue à l'article IV de la proposition de loi. L'Assemblée nationale à travers son rapporteur souhaite cette création pour 2 raisons un objectif pédagogique selon notre collègue député Erwan Balanant pour protéger, il faut définir un interdit fonction nécessaire à toute société est dévolu au code pénal. 2ème raison un objectif statistiques de suivi des plaintes pour harcèlement scolaire. Le Sénat partage ces objectifs d'ailleurs la rédaction que nous avions adopté en première lecture, permettait de réponse sur ces 2 points, la création d'une circonstance aggravante en cas de harcèlement d'un élève ou étudiant par l'un de ses pairs au sein d'un établissement d'enseignement, tels que proposés par nos collègues de la commission des lois permettant à la fois d'affaires mais un interdit clair, compréhensible par un mineur et de disposer de statistiques, j'ai pu le constater à l'occasion de l'audition de la Chancellerie par ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio dans le cadre des travaux préparatoires de premières lectures. La chancellerie a été en capacité de nous indiquer le nombre de dépôts de plainte pour harcèlement sur un mineur de 15 ans sur la 2ème, circonstance aggravante de l'actuel articles relatifs au harcèlement il y en a eu 35 en 2018, la chancellerie aurait été tout aussi capable de disposer de statistiques sur la circonstance aggravante de harcèlement commis sur un élève ou un étudiant par toute personne étudiants au sein du même établissement d'enseignement que nous proposions de créer le texte de l'article IV rétabli par l'Assemblée nationale durcit fortement les peines applicables, nous proposions une peine pouvant aller, selon les circonstances, jusqu'à 2 à 3 ans d'emprisonnement et 30 à 45000 euros d'amende d'amende en cas de harcèlement au sein d'un établissement scolaire, le texte de l'Assemblée nationale, prévoit des peines beaucoup plus lourdes de trois jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et de 45000 euros à 150000 euros d'amende. Quelle signification ont de telles quantum de peine pour des harceleurs qui sont dans la plupart des cas mineurs Thomas dessus la rappeler. Quel message pour les victimes et leurs familles lorsque les tribunaux n'appliqueront pas ce quantum de peine disproportionnée. La mission d'information alertait sur le risque de créer un tigre de papier avec ce délit spécifique, ce risque est d'autant plus fort avec des peines aussi élevé par ailleurs ce quantum de peine interroge profondément sur les ruptures d'égalité pour des faits aux conséquences similaires, le harcèlement commis sur un enfant lors d'activités périscolaires par ses camarades de club de sport ou encore par des jeunes de l'établissement scolaire voisin fréquentant les mêmes transports en commun au quotidien seraient donc moins punis pour des mêmes faits, commis par des élèves de son établissement scolaire. Pourquoi le cyber harcèlement sera-t-il plus grave lorsqu'il est réalisé par un jeune fréquentant le même établissement scolaire que la victime, même si le harceleur et le harceler ne se connaissent pas dans le monde réel, où est la cohérence lorsque l'incitation au suicide ou l'homicide involontaire sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende alors que les faits conduisant tôt suicide ou à la tentative de suicide en cas de harcèlement seraient commis serait pardon puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Quel message transmettre ces comparaisons en termes d'interdits sociétaux. Sur ces 2 points, définition du harcèlement scolaire : création d'un délit spécifique, le Sénat était ouvert un compromis en commission mixte paritaire. Malheureusement, ce n'était pas le cas de l'Assemblée nationale le rétablissement de son texte en témoigne j'en viens maintenant au cyber harcèlement dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre, nous avons enrichi le texte en première lecture, afin que la prévention de la lutte, la prévention et la lutte contre le SIDA, harcèlement soit spécifiquement mentionné dans le texte au moment de la formation initiale et continue dans les mesures que doivent prendre les établissements scolaires face à ce fléau ou encore ou encore lors de l'information annuelle délivré aux élèves et aux familles. L'Assemblée nationale a supprimé toute mention du cyber harcèlement sauf à l'occasion de cette sensibilisation annuelle des élèves et parents d'élèves. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale mentionné le cyber-harcèlement aux côtés du harcèlement scolaire serait davantage une source de confusion que de sécurité pour les élèves. Toutes celles et ceux qui ont participé à la mission d'information. On aboutit à la conclusion contraire je ne partage pas du tout ce point de vue, la mission sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le SIDA, harcèlement, a montré combien il était urgent de s'attaquer à ce problème, vous avez commencé à le faire, je le ministre notamment avec cette application dont vous nous avez parlé.

En outre ce cyber-harcèlement il se diffuse désormais dans le primaire, avec l'abaissement de l'âge de possession du 1er smartphone et d'inscription sur les réseaux sociaux. Ne pas faire référence au cyber harcèlement dans un texte qui se veut pédagogique, c'est minorer une réalité. Je m'interroge également sur la rédaction de l'Assemblée nationale qui limite la mention du cyber harcèlement à cette information annuelle des parents et des élèves. Comme si cela relève uniquement de la sphère privée et ne concerne pas l'institution scolaire. Les travaux de la mission d'information était pourtant explicite, je cite : ce serait une erreur de penser que le cyber harcèlement n'a pas de lien avec l'institution scolaire et ne doit donc pas être combattue par l'école. La mission sénatoriale appelait également au développement d'un savoir-être plutôt que d'un savoir-faire rapidement obsolètes en raison de la course constante aux innovations techniques et à l'émergence de nouveaux réseaux sociaux, cela concerne les parents et les élèves, mais aussi tout le personnel de l'Éducation nationale. Hasard du calendrier, je viens de le dire mais la semaine où l'Assemblée nationale minoré la mention du cyber harcèlement de steacks vous annonciez. Depuis, un établissement scolaire, le lancement de cette application dans le cadre du Safe Internet dès préféré que ce soit en français, avec pour but de faire en sorte que chaque élève puisse signaler un cyber harcèlement harcèlement scolaire et cyber-harcèlement sont présentés côte à côte dans vos déclarations, monsieur le Ministre, il est regrettable que ce soit trop peu le cas dans ce texte et nous avions décidé, nous au Sénat que le mot cyber harcèlement devait se trouver dans le titre même de la proposition de loi d'autres dispositions d'autres rétablissement pardon de dispositions de l'Assemblée nationale en ouvert les lectures sont regrettables, je pense à la création d'une nouvelle mission pour le réseau des Oeuvres universitaires notre alerte sur son financement n'a malheureusement pas été entendu les désaccords sont persistants et porte sur des dispositions majeures du fait du rétablissement par nos collègues députés de leur texte sur ces points, la commission de la culture considère qu'un nouvel examen détaillé de la proposition de loi ne permettrait pas de rapprocher les points de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer la commission propose à la haute assemblée d'adopter la présente motion tendant à opposer la création, la question préalable sur ce texte, je vous remercie.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en soutenant cette question préalable notre groupe formalisent l'expression d'une ambition déçue et non d'une obstruction car jamais l'obstruction n'a été dans l'ADN du Sénat, et encore moi sur ce texte, il est à cet égard tout à fait regrettable que la CNP du 1er février n'aient pas abouti, alors que le Sénat s'inspirant des contributions de sa mission d'information a enrichi le texte dans un souci d'efficacité in fine est l'une des seules avancées substantielles conservés dans le texte final concerne les assistants d'éducation, acteur incontournable de la lutte contre le harcèlement scolaire qui se voient proposer un CDI au terme de leur engagement contractuel de 6 ans mais le texte issu de la 2ème lecture ne prend pas suffisamment en compte le cyber harcèlement son effet son effacement sémantique et très mauvais est un très mauvais signal envoyé, surtout au regard de la réalité des chiffres quand nous savons que 73 % des moins de 13 ans possèdent un compte sur un réseau social et que 9932 procédures pénales ont été ouvertes pour des mineurs victimes des faits commis sur internet mais pire encore, mes chers collègues, au risque de me répéter ce texte instead une définition du harcèlement scolaire potentiellement ravageuses pour l'autorité du maître maître et du professeur, comment comprendre que sur la caractérisation même de ce mal la 1ère chambre s'faire dans une posture au détriment de la sécurité des adultes, enseignants, comment tolérer dans dans un contexte, hélas, marquée par un mouvement de SAP, de toute autorité, l'ouverture d'une telle brèche dans une institution scolaire dont l'autorité s'effrite chaque jour davantage l'inclusion dans la définition de l'harcèlement scolaire des faits commis sur sur un enfant par un adulte n'est ni juste ni pertinente, car elle ouvre la voie à d'irrémédiables abus des abus qui noir, on les voit des vraies victimes dans un ballet de dénonciation hasardeuses et qui empêcheront d'agir les garants de l'autorité, qui sont pourtant le seul salut des victimes, nous ne votons donc pas cette question préalable dans un esprit chagrin polémique ou vindicatif mais devant l'impasse habilité de la deuxième lecture, il nous fallait faire preuve de responsabilité, il n'est plus l'heure d'étendre nos discussions car ce texte quoiqu'imparfait doit entrer en vigueur au plus vite son avènement aurait été d'autant plus grands dans l'absolu consensus de mon cher collègue, vous ne l'avez pas permis Monsieur le Ministre, dont acte. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais rappeler les réserves que j'ai exprimée lors de la discussion générale concernant d'une part la la la reconnaissance du cyber harcèlement le harcèlement et je rejoins par là, le rapporteur de la commission, le cyber-harcèlement est extrêmement important important dans l'affaire qui nous préoccupe, c'est de nos jours le sujet le plus important parce que l'enfant qui est harcelé à l'école va continuer à l'être, via son smartphone ou sa tablette lorsqu'il rentrera chez lui, et là il y a vraiment un problème majeur, donc le fait que le le le nos collègues de l'Assemblée nationale n'est pas accepté que si cyber harcèlement soit mentionné est extrêmement grave, d'autre part, la demande de création d'un délit spécifique n'est pas tout à fait conforme avec les conclusions de la mission d'information sénatoriale, je rappelle que le triptyque : prévenir, détecter traité sur lequel le rapport de la mission s'est appuyé était vraiment au coeur de notre de nos, de nos travaux, en dépit de ses réserves, le groupe votera contre la mission, la question préalable parce que bon, d'une façon générale, nous sommes contre les questions préalables parce qu'on s'arrête de débattre, parce que bon c'est vraiment laissé une discussion en l'état, alors que le sujet mérité de d'avancer et de trouver des moyens d'action pour lutter contre le harcèlement scolaire et cela, je le regrette, donc, nous voterons contre. Merci, cher collègue Madame brûlant. Merci monsieur le président, notre groupe votera pour cette motion tendant à opposer la question préalable. En m'interrogeant et plus nous avançons dans ce débat, plus je suis interrogatif sur les raisons qui n'ont pas permis que cette CMP soit conclusive et si vous m'y autorisez monsieur le ministre, votre refus d'argumenter, votre avis défavorable, ce qui n'est absolument pas dans vos habitudes pour nous tous qui vous connaissons désormais bien me laisse encore plus interrogative sur les motivations profondes qui ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui, parce que je crois que nous l'avons encore montré aujourd'hui personne ici n'ignore le fléau. Qu'est le harcèlement plus encore à l'heure est à l'ère des réseaux sociaux des plateformes qui font que des enfants, des jeunes non plus un instant de répit, lorsqu'ils sont confrontés à cette situation qui conduit, on le sait, à des drames, mais la question qui nous est posée à tous, c'est comment lutter efficacement contre ce phénomène qu'il y a des des des implications extrêmement diverses, des causes multiples et qui nécessitent qu'on les traite, dans leur diversité et dans l'ensemble des aspects qu'elle recouvre, je crois que rien ne s'opposait véritablement à ce que ce travail soit fait, il y a eu des propositions constructives travailler ici au Sénat, il y en a eu aussi à l'Assemblée, et je pense qu'on pouvait tout à fait trouver le chemin d'un consensus que ça aurait été de bon augure que nous montrions ce visage à l'ensemble de la société et à l'ensemble de la communauté éducative et des jeunes, et encore une fois, pour des raisons obscures, ça n'a pas été possible, je le regrette profondément, voilà pourquoi nous voterons cette motion. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur. Monsieur le président. vraiment dans le prolongement de la mission madame et de Madame, Mellow et qu'on a vraiment, je crois, étayer nos positions de manière extrêmement forte on s'est même inspiré, Monsieur le Ministre, tout ce que vous avez pu dire lors des débats sur le projet de loi sur l'école de la confiance, et lorsque la question avait été abordée, nous avons pu constater, et nous le regrettons, sur un sujet aussi important, l'impossibilité d'ouvrir le dialogue. Avec nos collègues de l'Assemblée nationale dans la position nous a surpris sur ce texte, sur lequel nous aurions pu arriver à un consensus l'les rapporteurs étaient prêts à entrer dans une discussion sur un sujet qui méritait de consensus, mais nous avons eu par trop l'impression que le texte d'AscendEX était à prendre ainsi. Et cela explique que la commission soit ici positionné ce que je regrette ce que nous regrettons profondément. Merci, monsieur le rapporteur oui courte intervention. Serez-vous, je serai très bref, simplement pour regretter l'issue de ce débat, mais remercier très sincèrement, celles et ceux qui ont pris part, non pas seulement aujourd'hui mais, dans les précédentes journées de débats pour la qualité et la sincérité de leur engagement et exprimé pour terminer quand même un grand regret : Monsieur le Ministre, le regret de ne pas avoir entendu votre position sur cette question du harcèlement entre pairs, nous avons entendu votre position en 2019, mon petit doigt me dit qu'elle a pas vraiment changé et le fait que vous n'ayez pas osé répondre tout à l'heure. Comme l'a dit Madame Brulin est quand même très gênant le 1000000 de personnes qui travaillent pour l'éducation nationale qu'qui soient, professeur, qu'ils soient médecins scolaires qui soient ESH qui soit vs. Ils sont stigmatisés, d'une façon certaine par cet article 1 et le message que vous leur envoyez par votre silence. Me surprend beaucoup, parce que nous connaissons tous votre engagement pour soutenir. Les enseignants, le monde enseignant et je suis vraiment très navré parce que je pense que vous êtes malheureux aujourd'hui. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez tout fait pour me faire parler, là, donc je ne voudrais pas vous décevoir une seule fois en un quinquennat donc je vais évidemment vous répondent parce qu'on ne peut pas toujours dans les débats parlementaires s'exprimer, à chaque fois de serait ce que parce que le la présidence pourrait s'en inquiéter le à chaque fois que vous même que vous inquiéter d'un éventuel silence j'ai toujours répondu et je ferai pas exception aujourd'hui, donc je ne vais pas rester silencieux et je ne vais évidemment pas non plus de ce que vous avez entendu tout à l'heure à la tribune, ni de, de, de la compréhension qu'on peut avoir de mon avis défavorable, je voudrais d'abord dire que je comprends les débats qui ont eu lieu aujourd'hui, je veux dire il y a une noblesse de ce qui s'est dit il y a évidemment des arguments pour et contre ce parti, comme très souvent, heureusement dans dans les débats parlementaires et en fait on peut évidemment regretter, comme à chaque fois que ça se passe, le fait que les 2 assemblées n'ait pas pu s'entendre mais il y a évidemment de part et d'autre des arguments importants, pourquoi cet article, on en comprend l'inspiration, c'est de permettre vraiment de lutter contre le harcèlement dans tous les cas de figure qui existe et il est exact que dans le passé des faits divers. Peuvent correspondre à ce que vise cet article et pourquoi votre position si je veux la résumer, vous redoutez et je le comprends, aussi les effets pervers et le fait de mettre, le cas échéant des adultes, pas seulement les professeurs d'ailleurs dans une situation qui irait dans le sens d'ailleurs d'une judiciarisation excessive de la de la vie scolaire, qui est aussi une chose contre laquelle contre laquelle je je mets en garde donc les 2 positions sont des arguments tout à fait défendable, ce qui je regrette moi aussi que il n'y a pas eu la possibilité de la part de tout le monde, de trouver un un terrain d'entente, puisque ce terrain d'entente aurait pu aussi permettre que certaines choses comme la distinction effectivement trop harcèlement et cyber harcèlement que vous avez évoquées puis être davantage ancré, ceci n'est pas si grave, puisque, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure monsieur le rapporteur, cette distinction, elle est faite de toutes les façons, par le ministère de l'éducation nationale dans son travail et donc le débat est plus théorique qu'autre chose sur ce point, puisque évidemment que le cyber-harcèlement est compris dans le harcèlement et évidemment que nous prenons à bras le corps le sujet du du cyber harcèlement donc ce qui est très important, c'est d'abord de mettre en regard cette nouvelle disposition avec d'autres dispositions protectrices des professeurs et que j'ai souhaité et qui existe, je rappelle que l'article 1 de la loi pour l'école de la confiance qui, évidemment, reste en vigueur, comporte notamment dans sa 2ème phrase quelque chose qui est protecteur des enseignants et notamment contre évidemment toute dénonciation calomnieuse et contre toute autre problème il y a des déclarations que j'ai fait et qui reste valable, et qui se sont traduites dans des textes comme celui-là, et qui est que, évidemment, que la parole du professeur est fondamental qu'elle ne saurait être prise comme une parole, je dirais, de, de, de même nature que celle qui serait celle d'un d'un élève et évidemment qu'on ne qualifie pas de harcèlement n'importe où, n'importe quoi, ce qui était important c'est aussi évidemment la sagesse dans la mise en oeuvre des dispositions y compris celles qui pourraient avoir un caractère réglementaire dans dans dans les temps qui viennent, donc je ne dévie pas d'un centimètre sur le fait que nous devons la protection à nos professeurs et à l'ensemble des adultes qui travaillent pour l'éducation qu'il relève de la fonction publique d'État ou de celle des collectivités territoriales, que ce texte en aucun cas ne doit déboucher sur le sur une fragilisation juridique de la situation des des professeurs que nous pouvons pour cela compter à la fois sur l'équilibre que proposer que permettent les autres textes sur évidemment les dispositions réglementaires d'accompagnement. Et sur le fait que le 15 et, le cas échéant sur la sagesse des acteurs, y compris d'ailleurs le le le le juge dans dans l'école et dans les cas les plus extrêmes, mais en même temps, il y aura un progrès pour les cas justement extrême où cette disposition permettra d'avoir le l'angle large je peux comprendre ce certaines des interventions, elle me semble inspirée par une approche par les effets pervers et après tout ce n'est pas une approche aberrante parce qu'il faut en effet éviter les, les, les effets pervers, mais on peut aussi contenir les effets pervers et c'est évidemment ce que tout le monde fera, à commencer par moi-même, au travers de tout ceux qui accompagnera cette loi, je vous remercie. je vous rappelle que l'avis de la commission favorable, l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin 105 sur la motion, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politique et la présidence nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 342 pour l'adoption 214 contre 128 le Sénat a adopté cette motion donc le texte n'est pas adopté. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle Examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône. La parole est à monsieur Patrick Chauvet, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire pour 5 minutes. Monsieur le président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône est parvenu à un accord, je me félicite que le Sénat et l'Assemblée nationale soit convenu d'un compromis sur un texte important pour prolonger, mais aussi pour sécuriser la concession du Rhône, attribué à la Compagnie nationale du Rhône, dite CNR. Preuve de cette importance, ce texte a été adopté à l'unanimité par le Sénat, c'est un signal très positif en direction de la CNR, acteur incontournable de la transition énergétique nationale et de l'aménagement du territoire rhodanien pour autant, il y a beaucoup à dire sur la méthode retenue par le gouvernement sur ce dossier, il aurait pu et dû prolonger par décret la concession de la CNR, sitôt les concertations préalables achevée par ailleurs si cette proposition de loi est salutaire pour la CNR étant donné le contentieux européen entourant les concessions hydroélectriques, elle ne résout pas les difficultés rencontrées par les autres concessions échues qui, faute d'être renouvelé. Ont été placés sous le régime des délais glissants 39 concessions sur un total de 400 soit 10 % relève de ce régime. Le gouvernement doit enfin proposer une solution globale, concrète et négocier afin de sortir par le haut de cette situation d'insécurité juridique sans rien sacrifier de notre souveraineté économique ni de notre transition énergétique mais revenons sans à la proposition de loi lors de son examen au Sénat, nous avons veillé à inscrire la CNR sur la voie de la neutralité carbone en valorisant ses activités liées à l'hydrogène Vert et au photovoltaïque innovant, nous avons aussi voulu promouvoir le dialogue territorial en prévoyant la consultation des collectivités territoriales sur les projets de la concession dont un en suspens de 180 millions d'euros à Saint-Romain de et en garantissant leur éligibilité aux aides fournies par la CNR, nous avons aussi souhaité favoriser le développement agricole en prévoyant l'association du Ministre de l'Agriculture et en encourageant les emplois liés, il s'est agit en somme de fiabiliser de consolider le texte non d'en modifier l'équilibre général, le compromis de CNP a permis de conserver la totalité des apports sénatoriaux, c'est une grande satisfaction quelques ajustements mérite cependant d'être signalé tout d'abord, l'articulation entre le programme de travaux et le schéma directeur de la concession a été affinée de plus, l'autorité organisatrice de la consultation sur les modalités de réaffectations financières prévues en l'absence de réalisation du projet en suspens, a été précisée, il s'agit de la CNR pour les pour projet proposé et l'État pour les sommes réaffectés sur un autre point : la mission de soutien à l'emploi de la CNR a été étendue des emplois agricoles à ce locaux enfin la modification du cahier des charges et du schéma directeur a été autorisé par décret simple au total, l'examen du texte aura démontré tout l'intérêt du bicamérisme, sa rapidité pour prolonger la concession dans les meilleurs délais son utilité pour la garantir la sécurité juridique de cette prolongation je crois donc que nous avons fait oeuvre utile, c'est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement la présidente Sophie Primas le président Roland Lescure le rapporteur Patrick Monnier mignola toutes celles et ceux qui ont contribué à ce résultat et du travail fructueux qui a permis son aboutissement j'invite donc le Sénat a adopté le compromis de CNP, 100 ans après la loi de 1921 qui a fixé les missions historiques de la CNR il permettra la poursuite de la concession pour 18 années de plus et inscrira de surcroît ses missions dans les enjeux énergétiques et climatiques actuelles, je vous remercie. la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les les sénateurs, monsieur, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le le rapporteur, Monsieur le Sénateur Chauvet, merci, je suis à nouveau très honoré de de partager ce moment avec vous ce moment de de cohésion, si j'ose dire, autour de ce ce projet exceptionnel de cette structure, de cette CNR qui vraiment porte en elle cette compagnie nationale du Rhône, toute la promesse de ces enjeux que nous avons réconcilier enjeux économiques enjeux environnementaux enjeux sociaux énergétique nous trouvons autour de cette compagnie véritablement tous les tous les leviers et tous ce que nous avons à construire de ses équilibres à l'échelle d'un territoire entre ces différents enjeux enjeux agricoles aussi vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, puisque nous avons de cette gestion de l'eau à ce déploiement des énergies renouvelables à peu près tous les défis à l'oeuvre dans nos territoires, cette colonne vertébrale du Rhône 4ème fleuve européen le plus puissant de France sa biodiversité exceptionnelle, c'est 300 kilomètres de voies navigables son potentiel énergétique, on l'a dit, mais aussi, on le voit en termes de mobilité durable et notamment de transport fluvial font vraiment de ce de et de sept CNR l'âme du bassin rhodanien avec, nous l'avons vu une équipe, une équipe de près de 1400 salariés dont nous saluons aujourd'hui, le travail est vraiment l'engagement au coeur de s'territoire des énergies navigation une irrigation qui se développe également dans les énergies renouvelables, vous le savez, nous avons des enjeux extrêmement ambitieux dans notre mix énergétique de déploiement massif de ces énergies et au sein de de la Compagnie nationale du Rhône, nous trouvons à la fois évidemment l'hydroélectricité au coeur de ce projet, mais également le photovoltaïque demain sans doute, des projets qui montre puissance sur sur l'hydrogène et même l'innovation puisque dès 2023 la CNR démarrera un projet d'électricité osmotique, un projet pilote, au coeur de ces expérimentations aussi et de ses de cette recherche sur le déploiement de des énergies renouvelables, avec donc cette vision holistique si j'ose dire, à l'échelle du territoire et sur le temps long puisque cette prolongation que ce texte propose nous amène vraiment à à nous projeter s'était également une nécessité pour cette compagnie, comme pour les élus et collectivités de ce territoire que de pouvoir se projeter enfin et vraiment dessiner ses ses projets dans le dans le avec donc une prolongation que ce texte, vous propose de cette, de cette concession jusqu'au 31 décembre 2041 avec un texte que nous observons comme riche, équilibré et qui à la fois donc prolonge la concession mais aussi renforce les exigences de son cahier des charges et je crois que nous avons également trouvé une position de compromis et d'équilibre extrêmement appréciable la matière un texte également qui associe qui associe vraiment les différents acteurs sur ces 27 hectares sur ces 3 régions c'est 11 départements français, nous avons une centaine de collectivités actionnaires et une présence aujourd'hui de tous les niveaux de de collectivités, tous les acteurs autour de ce de ce projet, qui seront associés vraiment aux réflexions avec avec les élus, alors je souhaite vraiment à nouveau salué l'esprit de consensus qui a présidé assez à ces travaux parlementaires vous remercie à nouveau monsieur le rapporteur, madame la présidente pour le le travail récent jusqu'à 7, cette commission mixte paritaire conclusive qui nous permet d'espérer aujourd'hui une belle unanimité qui a été trouvé en en première lecture, déjà dans les 2 chambres remercier bien évidemment Patrick Mignola qui est l'auteur de cette proposition de loi et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et et vous dire à quel point j'ai été honoré de de participer à la prolongation de cette, de cette et d'observer cette mobilisation de la représentation nationale, qui est vraiment une belle reconnaissance je crois pour tous les porteurs et ceux qui font vivre ce projet de la Compagnie nationale du Rhône, et aussi la preuve que les bons projets Les projets forts les projets ambitieux et nécessaire ça veut trouver un beau consensus et s'affranchir merci à tous, évidemment, vous l'aurez compris le gouvernement soutient pleinement l'adoption de cette proposition de loi, je vous en remercie. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat statut par un seul vote sur l'ensemble du texte nous passons aux explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 5 minutes. Monsieur le président. Madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi afin d'examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue à un accord, il y a tout juste une semaine sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône ce texte d'initiative parlementaire, faut-il le rappeler, a pour objet principal de prolonger de moderniser la concession du Rhône, créé en 1921 et attribué à la Compagnie nationale du Rhône, la CNR qui est un modèle de concession unique en Europe, avant de revenir sur les principaux apports de ce texte, je tiens à remercier très chaleureusement, messieurs Patrick Mignola, auteur et rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale me joindre Madame la Ministre, aux souhaits de prompt rétablissement que vous lui avez souhaité et notre collègue Patrick Chauvel, rapporteur au Sénat pour leur investissement malgré des délais de travail contraint transition énergétique souveraineté énergétique, aménagement du territoire rhodaniens ont été les maîtres mots le fil rouge tout au long de l'examen de ce texte, c'est alors que, en tant que parlementaires de la Haute-Savoie, que je peux me réjouir que nos 2 chambres soient parvenues à un accord. Le Rhône ces 800 12 kilomètres c'est un fleuve qui prend sa source sa source dans le massif du Saint-Gothard en Suisse, au coeur d'un glacier qui traverse l'élément et qui parcourt toute la vallée qui porte son nom avant de se jeter dans le débat, dans le Delta de la Camargue dans la mer Méditerranée, dès 1921 la loi approuvant le programme d'aménagement du Rhône a fixé la à la concession, détenue par la Compagnie nationale du Rhône 3 missions historiques, la production d'hydroélectricité et l'irrigation agricole et la navigation fluviale, comme nous l'a rappelé, notre rapporteur Patrick Chauvet, il s'agit d'une entreprise remarquables en effet ces missions historiques, sa gouvernance mixte et son engagement sans faille en faveur de la transition énergétique font la Compagnie nationale du Rhône, une entreprise annule pareil et j'étais assez celle dans mon département encore dimanche dernier, on voit les installations de cette compagnie sur le fleuve, les enjeux sont donc nombreux la concession attribuée à la CNR arrive à échéance en 2023, il était donc nécessaire que le législateur intervienne à défaut du gouvernement sinon cette concession aurait aurait été placé sous le régime transitoire dit des délais glissants, qui touche déjà 39 concessions hydroélectriques sur 400, soit à peu près 10 % mais aujourd'hui par ce texte que nous allons être amenés à voter dans quelques instants, il sera désormais inscrit dans le marbre de la loi que la prolongation de sa date d'échéance, ainsi que son cahier des charges générales s'étendrait s'étendront jusqu'en 2041, autrement dit la CNR reste à l'abri du contentieux européen au moins pour quelques années encore, les accords, les apports du Sénat et les 4 axes qui avaient été définies ont été sauvegardés pour rappel : il s'agit du développement des énergies renouvelables, d'une meilleure intégration des collectivités territoriales, quant aux prises de décisions du comité de suivi de l'exécution de la concession, un seul chiffre, ce ne sont pas moins de 183 collectivités qui sont adhérentes à la concession du soutien aux professionnels agricoles et enfin du renforcement de la sécurité juridique de la concession, la commission procéder simplement à quelques ajustement rédactionnels et de bon sens ainsi l'articulation entre le programme de travaux et le schéma directeur a été précisée, s'agissant des modalités de réaffectations financières prévues en l'absence de réalisation d'un projet hydroélectrique hydro-électrique en suspens, pardon, l'autorité que ce soit la CNR où l'État procédant à cette consultation a été ajustée ou encore dans l'émission de la CNR ont été promus les employes locaux au côté des emplois agricoles des apports substantiels donc qui renforce juridiquement, le texte, mes chers collègues, vous l'aurez donc compris il était était impératif que le législateur s'emparent de cette problématique du prolongement de la CNR afin qu'elles ne passent pas sous le régime de la mise en concurrence, donnant lieu à un contentieux avec la Commission européenne aussi ce texte était très attendue par les îles locaux afin de d'appréhender au mieux les différents travaux à venir sur sur leur territoire, projet de barrage d'écluses, etc, c'est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe de l'Union centriste soutiendrons et voterons en faveur de la rédaction, établie par la commission mixte paritaire, sur cette proposition de loi merci. dans la suite de la discussion. La parole est à monsieur Bernard Fiolet pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi nous offrent l'occasion rare de nos prolongée sur le prolongement d'une concession hydroélectrique sans mise en concurrence, la concession d'aménagement du Rhône octroyée au concessionnaire actuel depuis 1934 qui fournit tout de même un quart de la production hydro-hydraulique de notre pays, cela est d'autant plus exceptionnel que l'accord préalable des services de la Commission européenne a pu être obtenue en l'espèce. Comme l'avait souligné Édouard Herriot en février 1946 il est plus facile de construire un barrage en Pierre ou en béton que de forcer les barrages des bureaux. N'est-ce pas. La situation singulière du concessionnaire, la Compagnie nationale du Rhône explique la relative facilité avec laquelle la France a pu obtenir sa prolongation pour 18 années supplémentaires, soit jusqu'en 2041, cela a été rappelé à maintes reprises la CNR a été privé de l'exploitation des barrages de 42 19146 à 2006 en raison de la nationalisation de la production de l'énergie. Que le Parlement puisse avoir son mot à dire, alors que la prolongation de la concession d'aménagement du Rhône pouvait intervenir aisément par décret constitue à mon sens un point très positif toute consultation démocratique sur la politique énergétique de notre pays qui implique des engagements de très long terme ne peut qu'être bénéfique, néanmoins, ne nous réjouissons pas trop vite sur l'avenir de notre Patrimoine hydraulique car nous ne sommes qu'à l'entrée du tunnel des contentieux en cours quant à l'application de la directive dite concession du 26 février 2014, rappelons-le, 150 concessions doivent arriver à échéance l'année prochaine. Une issue de préférence favorable à notre souveraineté énergétique doit être adoptée rapidement afin de déclencher une dynamique d'investissements dans un secteur clé pour la transition énergétique qui ne peut se passer de la houille blanche ainsi que ce que solutions de stockage de l'électricité, condition sine qua non pour atteinte l'objectif de 40 % de la part des énergies renouvelables dans notre mix électrique, les programmes pluriannuels quinquennaux apporteront ainsi 500 millions d'euros d'investissement. Outre sa mission relative à la production hydraulique, cette concession revêt également un caractère stratégique pour les territoires parcourus par le Rhône, que ce soit dans le domaine de la navigation fluviale ou l'agriculture, il convient d'être particulièrement vigilants quant à la gestion quantitative et qualitative de l'eau lorsque l'on sait l'enjeu que cela représente pour l'agriculture locale fortement dépendantes de l'irrigation. La prolongation accordée continuera donc de poursuivre les 3 missions historiques à l'origine de l'aménagement du Rhône, conformément à la volonté insuffler dès le départ. Comme cela avait été dit en première lecture par mon collègue Henri Cabanel la modernisation des contrats de concession doit être poursuivie dans l'ensemble des domaines d'intervention de l'État, notamment lorsque celle-ci nous engage pendant près d'un siècle, les prérogatives de puissance publique ne s'use que si l'on s'en sert point. Un État exigeant est un État concédant qui ne s'arrête pas à lire l'origine étymologique du mot concéder et qui ne se retire donc pas totalement de l'exécution du contrat. Qui ne doit pas entériner des situations acquises excessivement confortables pour le concessionnaire, comme on a pu le constater au sujet des sociétés concessionnaires autoroutières aussi l'insertion de clause de revoyure en 2028 2000 34 et la possibilité de modifier par décret le cahier des charges permettront, le cas échéant d'ajuster l'équilibre de la concession, cette souplesse est devenue plus que nécessaire. Concertation approfondie en amont, renforcement de l'association des élus à tous les stades de l'exécution de la concession durée raisonnable de la prolongation dans le cas de circonstances exceptionnelles, possibilité d'ajuster l'équilibre du contrat, les conditions nous semblent réunies pour maintenir le concessionnaire actuel dans son statut, la commission mixte paritaire à préserver les apports du Sénat, les modalités de la prolongation de la concession dans la proposition de loi sont favorables à la transition énergétique aussi le groupe RDSE votera en faveur de la présente proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est à madame. Florence Blain se comptant pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie, il y a quelques jours, sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône est parvenu à un accord et sénatrices et sénateurs, socialiste, écologiste et républicain se réjouissent que la CNR soit ainsi reconduite comme concessionnaire jusqu'au 31 décembre 2000 dans le texte qui nous est soumis, aujourd'hui, il apporte stabilité, sécurité et vision à long terme, à tous les professionnels et habitants des rives du Rhône, la présente proposition de loi reprend seul, a déjà été dit les 3 missions historiques de la CNR, à savoir la production d'électricité, le développement de la navigation sur le Rhône et l'irrigation pour l'agriculture, mais elle va plus loin en lui donnant les moyens d'être un acteur de la transition écologique, le changement climatique et ses effets s'impose à tous toutes nos politiques publiques doivent désormais le prendre en compte, c'est à la fois une contrainte, mais aussi une opportunité pour développer l'inventivité de nos chercheurs de nos entreprises, de nos services et la CNR a d'ores et déjà pris cette voie elle produit près d'un quart de l'hydroélectricité française, elle a aussi créé 49 parcs photovoltaïques et 57 parcs éoliens. Le texte que nous allons voter comporte en annexe un cahier des charges est un schéma directeur, il programme 500 millions d'euros d'investissement, dont 165 les 5 premières années, ils devront poursuivent les objectifs de la programmation pluri-annuelle de l'énergie et la neutralité carbone à l'horizon 2050 demeure de ce point de vue un objectif essentiel la prolongation de la concession de la CNR et la garantie d'une démarche de service au profit de tous et il est important pour nous et nous l'avons déjà souligné que cette société demeure sous contrôle public, en association avec les collectivités territoriales, que je le répète, la production électrique est un enjeu majeur pour lutter contre le réchauffement climatique et ça ne peut être conduit efficacement qu'avec une articulation forte avec les autorités publiques, qu'elle soit nationale ou locale. Dans le cas précis, nous avons contribué à renforcer le rôle du comité de suivi dans l'exécution de la concession, le Rhône traverse 3 régions, départements, avec 183 collectivités locales adhérentes et nous nous réjouissons également que les parlementaires soient associés à ce comité de suivi, outre la lutte contre le réchauffement climatique, les travaux programmés permettront de rénover et d'améliorer l'équipement de 6 barrages du Rhône et la continuité piscicole la CNR a pour mission de développer la navigation fluviale et de favoriser l'irrigation pour l'agriculture et, notamment, nous avons veillé dans ce texte, à maintenir un soutien aux employes issus de l'irrigation agricole et autres employes de la vallée du Rhône, élu du département de l'Ain, je serai évidemment très attentive à la consultation des différentes parties pour le projet, en amont du confluent de la à Saint-Romain déjà Leona et si ce projet ne pouvait aboutir à la réaffectation bien entendu des fonds. Au-delà de ce texte, je le souligne, c'est l'ensemble, et ça a déjà été dit par mes collègues, c'est l'ensemble du secteur hydroélectrique en France qu'il nous faut stabiliser pour l'avenir, je dois dire que pour l'heure, rien n'est fait, nous sommes dans une période où 10 % des concessions hydroélectriques sont arrivés à échéance, alors que le contentieux avec les institutions et la Commission européenne n'est en rien réglé, nous sommes donc dans la phase des délais glissant, dangereux pour ses concessions et je je souhaiterais que l'exécutif soit plus actif sur ce domaine pour traiter au fond le contentieux européen et pour sécuriser les autres concessions et installations hydroélectriques avec les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et réélu Publica, nous sommes très favorables bien entendu à l'adoption de cette loi, elle consolide un pan important de la production électrique en France, il s'agit maintenant d'oeuvrer pour qu'il en soit de même pour les autres concessions hydroélectriques et pour EDF, principal opérateur public du secteur, je vous remercie. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la cohabitation de l'homme de Néandertal avec l'Homo sapiens a été confirmée par des chercheurs, cela a été attestée par la présence de fossiles très par là dans la grotte de membres sur la commune de Malataverne dans la Drôme, à quelques kilomètres du Rhône, jeudi dernier, une telle découverte place ce fleuve comme un grand couloir de migration permettant à Homo sapiens de rejoindre l'espace méditerranéen et l'espace continental européen cette position stratégique peut s'expliquer par les brusques variations climatiques en Europe et en Asie, qui ont fait de notre fleuve Rhône un refuge climatique, vous me direz : quel est le lien entre les conclusions de notre CMP conclusive et ce qui nous réunit, ce matin, elle nous indique simplement que bien avant la Compagnie nationale du Rhône, l'espèce humaine a su tirer parti des ressources stratégiques de ce fleuve ces ressources aujourd'hui, économique et écologique judicieusement exploitée depuis un siècle par la CNR, cette dernière doit pouvoir continuer à les exploiter jusqu'en 2041 ce fut l'objet de notre courte commission mixte paritaire de jeudi dernier, de ces faits, nous rappellerons qu'il s'agit, depuis hier soir, de la 11ème CMP conclusive sur les 12 de nos 2 commissions, soit un taux de réussite de 92 ce qui démontre que l'apport législative du Sénat, hé bien pris en compte, je m'en réjouis, tout comme je me réjouis de la bonne entente de nos 2 présidents de commission Roland Lescure et Sophie Primas. Il faut dire que la Compagnie nationale du Rhône fait du bon travail et que la moindre des choses était de l'accompagner, et donc de s'accorder sur cette prolongation, je tiens à saluer ses représentants en tribune qui travaille particulièrement sur ce renouvellement de concession depuis 8 ans. Peu ou pas d'objection entre nos 2 rapporteurs sont à relever, bien au contraire, des modifications rédactionnelles de notre rapporteur Patrick Chauvet, que je remercie de son engagement, ont bien été prises en compte par l'Assemblée nationale, ces précisions permette de solidifier juridiquement, le texte, d'autres sont plus substantiel et permettent notamment aux territoires concernés d'être encore plus impliqués dans le processus de décision, je me félicite ainsi que le rapport annexé soit amendé pour que le comité de suivi émettre un avis sur les résultats des études relatives à l'éventuelle réalisation de nouvelle main d'un nouvel équipement hydroélectrique à singe crois Romain de ce projet suscite un certain nombre d'interrogations qu'il faut entendre, il conviendra d'être vigilant et constructif. Notre rapporteur a également veillé à inscrire la CNR sur la voie de la neutralité carbone en valorisant ses activités liées à l'hydrogène Vert et au photovoltaïque innovant des ajouts salutaire qui s'inscrit dans les engagements de la compagnie. Très innovantes dans la recherche de nouvelles opportunités pour favoriser la transition énergétique, la CNR a présenté en 2020, un parc photovoltaïque flottant au lac de la Madone, à quelques km de l'agglomération lyonnaise. Il s'agit de la première et unique plateforme en France, transversale, elle combine habilement irrigation énergie et biodiversité par l'État par l'installation de nurserie à poissons sous la plateforme et permis ainsi de concilier enjeux énergétiques et environnementaux. Par cet exemple, on comprend bien que la CNR est beaucoup plus qu'un seul concessionnaire pour la production d'électricité française nous démontre qu'il est tout à fait possible de bâtir un modèle économique qui produisent des richesses, donc de l'emploi sans gaspiller sans salir sans détruire, mais au contraire par les soeurs des énergies renouvelables et faire en sorte de notre territoire, un laboratoire pour l'invention de nouvelles ressources énergétiques, à présent, considérant que la CNR va pouvoir travailler sereinement à elle de nous démontrer que, dans les faits, ces actes, cet acteur clé de la transition énergétique pourra suivre les projets en faveur du développement et de l'équilibre des territoires au regard de ses actions et de la philosophie qui l'anime, elle conserve toute notre confiance et nous voterons bien sur ce texte en adressant tous nos voeux de prompt rétablissement Patrick Mignola lors de l'auteur de cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est au président Claude Malhuret pour les indépendants pour 5 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'unanimité est suffisamment rare pour être relevé cette proposition de loi la recueillis au sein des 2 chambres du Parlement, c'est dû à la fois au travail de compromis qui a été réalisé, mais aussi au sujet dont l'importance n'est plus à démontrer une nouvelle fois, je souhaite remercier notre rapporteur Patrick Chauvet pour son engagement sur ce texte. Et les précisions d'importance qui ont été apportées, je salue aussi le travail qui a été fourni par la Chambre haute, les modifications effectuées sont rigoureuses et équilibrée, peu de retouches ont été faites lors de la CMP, ce qui prouve que la qualité des échanges entrepris et les solutions envisagées en amont, hé bien là, comme j'ai pu le dire en première lecture le Rhône est un fleuve aux multiples atouts pour les territoires qu'il traverse et pour notre pays, soutenir et finaliser le prolongement de la concession de la Compagnie nationale du Rhône est primordial aux yeux de notre groupe, ainsi nous nous félicitons d'un accord rapide et pu voir le jour, le Rhône et plus largement les fleuves de notre pays constituent des opportunités en matière économique, industriel et écologique, la question des emplois en lien avec le fleuve et sur les territoires des départements, par lesquels il s'écoule en est le meilleur exemple le Rhône est vecteur de progrès. La France fait face à de nombreux enjeux, notamment celui de la lutte contre le dérèglement climatique, à ce titre, comme en première lecture, je me réjouis que le Sénat est inscrit dans la proposition de loi, l'aménagement du Rhône dans l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2005 cet aménagement est précieux pour les collectivités territoriales et les élus locaux protagonistes privilégiés et efficace des évolutions territoriale, il faut souligner le travail de coordination et les relations construites entre ces derniers et la Compagnie nationale du Rhône, le dialogue avec tous les acteurs en présence est synonyme de réussite pour les territoires et pour les Français, il doit se poursuivre et s'accentuer pour répondre au mieux aux enjeux actuels, c'est un exemple transposable pour d'autres territoires. L'aménagement du Rhône est aussi un formidable moyen pour répondre à l'objectif du développement du transport fluvial et la France se veut ambitieuse en ce domaine, cela participe à la décarbonation des transports, secteur très émetteur ou les solutions restent à financer et à inventer. La biodiversité est fortement impactée par la gestion des cours d'eau, l'Euro n'abrite une faune et une flore exceptionnelle la qualité de l'eau et l'aménagement sont 2 facteurs essentiels pour ces espèces, elles participent également à l'équilibre du fleuve. La qualité de l'eau et sa quantité suffisante sont un Avantage indéniable pour les cultures qui Borde le Rhône, les employes et les familles qui en dépendent, sont nombreux, chacun sur les territoires, a conscience que la bonne gestion du fleuve par la CNR est une nécessité, cela est d'autant plus vrai quand on en vient à l'hydroélectricité, j'avais déjà longuement appuyer mes propos sur ce volet la semaine dernière l'hydroélectricité constitue un espoir véritable concernant la production électrique et les objectifs de la PPE, le Rhône, il y a une place privilégiée car principal.

l'eau et l'énergie du présent comme elle sera celle de l'avenir. Les discussions au niveau européen, doivent se poursuivre, la France doit continuer à investir dans ce secteur, tout en préservant ses intérêts, cette proposition de loi propose une sécurité juridique adapté un cahier des charges est un schéma directeur au service des enjeux actuels multiple auxquels fait face le Rhône, elle est l'exemple d'un travail par le Menteur de qualité et de compromis, elles étaient nécessaires et les conclusions de la commission mixte paritaire, montre que l'exercice a été réussi pour toutes ces raisons, comme en première lecture, le groupe des indépendants votera à l'unanimité en faveur de son adoption. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Vivet Lopez pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord sur ce texte qui vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve du Rhône détenue par la Compagnie nationale du Rhône, je voudrais saluer à ce stade, le travail de notre cette assemblée et plus particulièrement celui de notre rapporteur Patrick Chauvet et de notre présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas depuis près de 90 ans, la CNR est un acteur incontournable de la transition énergétique, elle assure ainsi un quart de la production hydroélectrique dans notre pays et conduit des projets de recherche et d'innovation, particulièrement en matière d'hydrogène ou de photovoltaïque, la CNR est également un acteur majeur de l'aménagement du territoire rhodanien celui-ci comporte des aménagements variées comme des ouvrages hydroélectriques des sites industriels et portuaires, au terme de l'examen du texte, le territoire concédé se répartira sur 30000 hectares et 550 kilomètres de fleuves, seule la concession de QG géré par EDF et la traversée de Lyon géré par VNF et la métropole de Lyon demeureront hors du périmètre de la concession CNR le texte donne également une valeur législative au GAEC cahier des charges, général et au schéma directeur qui comprend un ensemble d'actions et d'objectifs Mian Oeuvres via des plans quinquennaux dont le montant atteint 165 millions d'euros pour le 1er et 500 millions d'euros au total, je me réjouis du programme de travaux supplémentaires pour, notamment, l'équipement de 6 barrages par des petites centrales hydroélectriques pour une étude de faisabilité d'un nouvel ouvrage hydro-électrique d'une puissance de 40 mégawatts dans le secteur de Saint-Romain De Gea pour une augmentation des capacités de production de l'aménagement hydroélectrique de Montélimar pour dépassa à poissons, ce texte est l'aboutissement des travaux et de concertations préalables et il y a débuté en 2019 à rien avec les élus locaux et les acteurs territoriaux tous soutiennent la prolongation de la concession, la Commission européenne a également confirmé la comptabilité de cette prolongation avait le droit européen, pour autant, le Sénat a souhaité enrichir le texte dans le sens de la transition énergétique du jazz, du dialogue territorial et du développement agricole, tout d'abord, développer les énergies renouvelables en plaçant l'émission de la CNR sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2050 un promouvoir les projets relatifs à l'hydrogène renouvelable au bac ou bas-carbone en soutenant l'utilisation de procéder photovoltaïque innovant ensuite associer les collectivités territoriales en territorialisant le comité de suivi de la concession en consolidant leur association à la lire, l'élaboration des programmes pluriannuels de travaux en consolidant leur consultations sur le programme de travaux supplémentaires et son état d'avancement, ainsi que sur l'évolution ultérieure du cahier des charges du schéma directeur et enfin soutenir les professionnels agricoles en première mieux en compte les emplois induits par l'irrigation agricole, dans l'émission de la CNR, en associant le ministère de l'agriculture au statut de la CNR et au comité de suivi de la concession en prévoyant que la compensation financière prévue pour les énergies réservé non attribué soit bien affecté aux actes, aux acteurs de terrain et non à l'État, la quasi-totalité des apports du Sénat ont été maintenus dans le texte issu de la CMP, c'est pourquoi le groupe Les Républicains votera pour le texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la justice. Si on la parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe Écologie Solidarité territoire pour 5 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe écologiste solidarité territoire soutient cette proposition de loi qui permet de reporter à 2041 la question de la mise en concurrence de la concession du Rhône qui arrive à son terme en 2023, un texte important qui prévoit la mise à jour du cahier des charges de cette concession et de son schéma directeur, permettant ainsi de moderniser les modalités et le périmètre d'activités cette actualisation prévoit, nous l'avons vu 500 millions d'euros d'investissement sur le Rhône, consacré à la production d'énergie hydraulique, le transport fluvial, l'irrigation ainsi qu'à des travaux environnementaux, dont 165 millions d'euros pour les 5 premières années avec un volet spécifique de 30 millions d'euros dédiée aux projets des collectivités locales, des mesures que nous saluons. Nous avons également soutenu en commission des affaires économiques, les apports du rapporteur, notamment la réaffirmation du cadre de transition énergétique, appelant à la neutralité carbone et le renforcement du dialogue territorial, nous aurions toutefois souhaité intégrer à ce cadre, la question de la préservation de la biodiversité qu'il est toujours utile de savoir rappeler et qui doit se concilier au déploiement de l'hydroélectricité, le Sénat a également contribué à rendre le texte juridiquement plus solide et a rappelé les objectifs nationaux de la programmation pluriannuelle de l'énergie, auquel la CNR doit pleinement contribuer. Nous nous félicitons de ces apports adopté au Sénat. Nous nous félicitons qu'ils aient été maintenus dans cette dernière version, mais si cette proposition de loi est utile et bénéfique pour la CNR, elle ne résout pas les problèmes majeurs de la mise en concurrence pour les autres concessions hydroélectriques, notamment celles qui sont détenues par le groupe EDF mise en concurrence imposés par 10 la directive européenne de libéralisation du marché de l'électricité 39 concessions hydroélectriques sur 400 sont arrivés à échéance et ont été placés sous le régime des délais glissants leur devenir et toujours très incertain et le gouvernement n'a toujours rien proposé comme solution pérenne. Le sélecteur de l'hydroélectricité attend des solutions globales concrète et négocier afin de sortir par le haut de cette situation d'insécurité juridique sans mettre à mal notre souveraineté économique ni notre transition énergétique. Avec le groupe écologiste à travers notre proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public, examiné en fin d'année dernière, la fin, la mise en place d'un véritable service public des énergies renouvelables, afin de répondre à à l'absence de politique publique efficace et apporter une vision stratégique sur ces questions majeures: un service public des énergies renouvelables permettrait d'amplifier notre transition énergétique de planifier de réguler le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays, d'accompagner les acteurs privés de structurer les filières industrielles et d'organiser la solidarité nationale permettant d'assurer un tarif unique de l'électricité partout en France, dans cette vision qui est la nôtre et nous l'avions déjà souligné lors de notre explications de vote, il est donc essentiel que la majorité des capitaux de la CNR demeure le statut hybride, mi-public, mi-privé de la CNR se posera d'ailleurs, à terme, c'est une garantie de stabilité, de perspectives à moyen terme pour l'entreprise et les salariés. Ce texte, que nous votons aujourd'hui est très attendue par les collectivités, les élus et les salariés, il est attendu aussi bien sûr pour notre politique énergétique, les enjeux climatiques et la biodiversité qui s'y rattachent. Il permet de mettre la CNR à l'abri du contentieux européen, c'est pourquoi nous nous voterons pour cette loi et resteront mobilisés sur ces enjeux majeurs de souveraineté de transition énergétique, je vous remercie. la parole est à Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 5 minutes.

mais aussi attendue pour les salariés qui, depuis 7 ans étaient dans l'expectative, c'est donc une issue positive qui nous réunit aujourd'hui et qui permettra à la compagnie nationale du Rhône de continuer d'oeuvrer pour les territoires de concert avec les acteurs locaux, il est utile de rappeler la CNR, ce sont 183 collectivités partenaires ce 50,3 % de capital issu du secteur public et pas moins de 14500 emplois Directs et indirects générés ont vallée du Rhône, notamment grâce à une politique d'achat concentrés à 85 % sur des entreprises locales. La CNR montre son statut d'entreprise structurante du territoire, et il faut se féliciter que cela continue pour de nombreuses années en étant le 1er producteur d'énergie exclusivement renouvelable en France, la CNR s'inscrit parfaitement dans la politique de lutte contre le changement climatique. Avec ses 19 barrages et ses 49 centrales hydroélectriques, elle produit 25 % de l'hydroélectricité française petit aparté, je veux tout de même rappeler ce que m'a dit ma collègue Cécile Cukierman, en première lecture sur le développement de l'hydrogène, je veux insister sur le fait que ce développement nécessitera des besoins en eau supplémentaire, tout comme le maintien, voire le développement du parc nucléaire, nous devons donc travailler à cette sécurisation en nous, respectueuse de l'environnement, faisant travailler localement nos concitoyens : il ne manquerait plus qu'elle soit rentable pour l'ériger en modèle qui fonctionne, hé bien c'est le cas. Puisque la CNR est aussi extrêmement rentable, avec un chiffre d'affaires d'un milliard et demi et un résultat Net se situant entre 90 et 100 millions d'euros, sans vouloir faire de digressions trop importante, je veux simplement rappeler au gouvernement qu'EDF, c'est un résultat Net de 650 millions d'euros et qu'Aeroports de Paris, avant la crise Covid c'était un résultat Net de 588 millions d'euros, à capitaux majoritairement publics sont donc très souvent excédentaire, ne les laissons pas à la main des grands groupes privés comme nous l'avons fait pour les autoroutes, pour lesquels nous nous Bourdon aujourd'hui les doigts madame la Ministre, je vous le dis, notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins, les décisions qui seront prises dans le dossier EDF peuvent être lourde de conséquences pour notre nt énergétique sur la lutte contre le réchauffement climatique mais également sur l'emploi liées à l'industrie électrique dans notre pays, l'État le gouvernement doivent être en capacité d'apporter une réponse cohérente qui montre qu'une autre voie que celle de la rentabilité peut exister, nous devons être guidé par une démarche qui répond aux besoins des Françaises et des Français de nos entreprises et à la décarbonation de la consommation énergétique, je fais le voeu que l'adoption de cette proposition de loi. Dans l'unanimité et je salue le travail de notre rapporteure soit le point de départ d'une nouvelle façon de concevoir le service public de l'énergie, celle de le voir comme un bien commun, or je le redis ici un bien commun ne peut en aucun cas être libéralisée, le simple fait que l'énergie soit pensé comme un service public implique qu'il soit sorti des logiques de concurrence et de marché, respectueux de l'environnement et au service de la population des territoires, je souhaite sincèrement que le modèle de la CNR soient à l'esprit de chacune et chacun, si toutefois, dans les mois et années à venir, nous devrions examiner un énième texte visant à privatiser nos services publics et comme tout le monde le sait évidemment, nous savons que si vous nous faites un second mandat, nous aurons le projet recule mais évidemment si telle était le cas, nous saurions face à vous, pour contrecarrer ce projet, je vous remercie. Merci, cher collègue. Alors, conformément à l'article 42 Alina 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans La rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

remercier les rapporteurs, le gouvernement et dire qu'effectivement cher Fabien nous faisons oeuvre utile mais je ne voudrais pas que nous finissions d'examiner ce texte, c'est tout nouveau votions se rendre hommage au travail d'Élisabeth Ayrault dans les années précédentes, qui a dirigé la CNR présidé la CNR et je voudrais remercier remercier souhaiter le meilleur à à sa nouvelle présidente, Madame Boroumand, celle qui est dans les gradins et dire à toute l'équipe de la CNR, que le Parlement dans son entier donne toute notre confiance, toute sa confiance à l'ensemble de l'équipe CNR pour continuer l'oeuvre utile qu'ils font sur ce fleuve. Merci madame la présidente.

Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. La parole est à Monsieur Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour 5 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, Sophie Primas, mes chers collègues. Je suis particulièrement heureux de soumettre aujourd'hui à votre vote le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur qui s'est tenue le jeudi 3 février dernier. Les débats entre les 2 chambres ont été vifs animé mais ils ont permis d'aboutir à de très nombreux compromis utiles et consensuelle, sur un sujet auquel font face, la majorité de nos concitoyens au moins une fois dans leur vie. Je pense qu'elle est ce qu'avec ce texte, nous mettons un point final à une aventure l'initiative qui dure depuis une dizaine d'années qu'il aura non seulement permis l'ouverture à la concurrence de ce marché, mais également grâce aux travaux nos chambres de grandes avancées en matière de justice sociale. Je me réjouis donc que nos 2 chambres se soient entendus pour avancer sur ces sujets, je voudrais là aussi saluer ici le travail de l'écoute. Et surtout du temps qu'on a, on a passé ensemble à essayer de construire ce compromis de avec notre ma collègue rapporteur de l'Assemblée nationale, Patricia Lemoine. Je voudrais la remercier et remercier toute son équipe, parce qu'effectivement, nous avons passé avec notre équipe et je voudrais remercier aussi Laurent et Sébastien à mes côtés et, bien sûr, avec le soutien de notre présidente effectivement c'était pas simple, on est parti de loin. Et on est parti de loin, même dans un contexte où il y a eu tellement de mensonges, de 10 par certaines associations, qui d'ailleurs était très parfois liées à des alternatives. Mais ce qui est important aujourd'hui, mes chers collègues, monsieur le ministre. C'est que, vous le savez, nous avions refusé en première lecture, de faire le pas même Paris, que l'Assemblée nationale concernant la réalisation à tout moment l'honnêteté m'oblige à redire que nous pensons qu'elle n'apportera quasiment aucun gain aux consommateurs, mais qu'elle représente plusieurs risques, notamment celui de la démutualisation qui pénalisera en priorité les publics les plus vos âgés et les plus fragiles, toutefois, le compromis que nous avons trouvé qui reprend la quasi-totalité des apports du Sénat sur le volet médical rend ce pari plus acceptable la protection que nous apportons au public vulnérable, frappé par la maladie ou l'ayant été et significative dès lors et à condition que l'information du consommateur soit grandement renforcé et nous est apparu légitime de valider cette disposition de la proposition de loi. J'en viens maintenant au contenu du compromis, comme indiqué à l'instant, l'article 1er permettra désormais de résilier son assurance emprunteur à tout moment. Alors qu'il fallait jusqu'à présent, respecter certains délais mais compte tenu de l'inutilité d'un droit de résiliation si les consommateurs ne le connaissent pas le Sénat, a été entendu sur son souhait que les assureurs informe désormais chaque année les assurés de ce droit et de ses modalités de mise en oeuvre nos travaux sur le renforcement des motivations des décisions de refus des prêteurs sont également conservés de même les articles additionnels que nous avions introduit et qui participent du rééquilibrage du rapport de force entre l'emprunteur et le prêteur sont maintenus et sera donc interdit pour un prêteur de modifier le mode d'amortissement d'un prêt et devra afficher le coût de l'assurance emprunteur sur 8 ans. Mais le plus important. Le travail de nos 2 assemblées se sont en effet mis d'accord pour conserver la quasi-intégralité de nos travaux sur le droit de l'oubli à l'oubli et sur la suppression du questionnaire médical dans le détail, le droit à l'oubli, réduit de 5 de 10 ans à 5 ans pour les pathologies cancéreuses et l'hépatite C par ailleurs la convention Heras travailler sur un élargissement de ses droits et de sa grille de référence à de nouvelles pathologies notamment chronique en l'absence de résultats il est exigé du gouvernement qu'ils agissent avant le 31 juillet 2022 questionnaire médical, quant à lui, reste supprimée pour les prêts de moins de 200000 euros par personne, soit 400000 euros pour un couple, et sous réserve qu'il ne se termine avant les 60 ans de rassurer, nous avons également prévu qu'un décret puisse faire évoluer ces seuils, oui, mais uniquement dans un sens plus favorable pour l'emprunteur, mes chers collègues, j'imagine que c'est également le cas pour vous mais je tiens à souligner le nombre de courriers de remerciement, j'ai reçu sur ce sujet de la part de concitoyens qui m'indique que c'est la fin d'un cauchemar : la fin d'un cauchemar de plusieurs années pour eux, nous avons fait oeuvre utile et nous pouvons être fiers je tiens aussi à préciser que le risque de hausse soudaine des tarifs brandies par certains assureurs n'est pas crédible parce que nous avons renforcé la concurrence je voudrais tout simplement à cet instant, vous dire que ce texte de loi, en plus c'est un texte vivant puisque par simple décret, vous pourrez me quel que soit le gouvernement, augmenter le niveau des 200000 euros, augmenter l'âge des 60 ans par un simple décret par le travail de la convention Area on pourra tout simplement aussi, j'ai terminé président je vous rassure. On pourra tout simplement aussi exclure de nouvelles pathologies chroniques qui perd Bertrand attendent famille construire acheter une maison, acheter un appartement, c'est souvent un projet de vie, je voudrais vraiment vous remercier

Monsieur le ministre, Olivier Dussopt ministre délégué, chargé, chargé des comptes publics. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, suis très heureux d'être devant vous pour évoquer et adopté cet après-midi, je le souhaite, des conclusions de la commission mixte paritaire portant sur la proposition de loi portée par la députée Patricia Lemoine et qui vise à garantir un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché l'assurance emprunteur, cette proposition de loi représente un véritable gain de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, la possibilité de changer à tout moment, ce contrat d'assurance va permettre aux Français de gagner environ 550 millions d'euros de pouvoir d'achat par an et, ainsi, un je ne contractants pardon, un emprunt pour acquérir, pour la première fois, sans logement pourra choisir de changer à tout moment d'assurance et ainsi en moyenne plus de 3800 euros sur la durée de ce prêt, cette mesure a un autre mérite aux yeux du ministre du Budget, je suis, c'est une mesure qui ne coûte pas un Euro à l'État, c'est une simplification sont des droits nouveaux pour les emprunteurs, sans que cela Vienne grever les caisses de l'État, l'accession à la propriété, représente pour beaucoup de nos concitoyens, vous le savez, l'objectif de toute une vie, il repose essentiellement sur le crédit immobilier qui est lui aussi très souvent conditionnés à la souscription d'une assurance emprunteur cette assurance peut parfois représenter jusqu'à 30 % du coût total du crédit, ainsi l'accès d'une accessibilité d'une assurance emprunteur au meilleur prix, confortant de pouvoir d'achat des Français est évidemment une préoccupation phare du gouvernement, la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui répond à 2 objectifs essentiels que le gouvernement soutient bien évidemment d'une part, elle vise à permettre aux Français de changer à tout moment son contrat d'assurance afin de garantir un libre choix et la possibilité pour chacune et chacun de bénéficier de meilleures garanties, et ce au meilleur tarif, et d'autre part, cette proposition de loi permet de réduire les discriminations d'accès des personnes atteintes ou ayant été atteintes par des maladies de longue durée, c'est aussi une question de justice sociale devant l'accès à la propriété et l'accès au propre et qui le conditionne le marché de l'assurance emprunteur compte entre 20 et 25 millions de contrats actifs et au cours de la dernière décennie, le législateur s'est légitimement pencher à plusieurs reprises sur ce sujet pour que l'assurance emprunteur protège les assurés à un coût qui sera le plus compétitif, les réformes qui se sont succédé depuis 2010 ont d'ores et déjà permis des avancées significatives, le marché de l'assurance emprunteur pour le crédit immobilier s'est progressivement ouvert à la concurrence, chacun devait avant 2010 adhérer au contrat de groupe qui pouvait lui être imposées par sa banque les emprunteurs ont aujourd'hui de tout le loisir de retenir l'assureur de leur choix est un choix qui est désormais n'est plus irrévocable de plus la possibilité de résilier son contrat est possible à tout moment jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, puis lors de chaque échéance annuelle, c'est cet aspect du droit que cette proposition de loi va pouvoir améliorer ses réformes depuis 2010 ont faciliter le changement d'emprunteurs et ont déjà offert des bénéfices substantiels pour les consommateurs, pressions des précédentes réformes mettent en évidence un renforcement de la concurrence et une baisse de la tarification des contrats d'assurance emprunteur, pour le plus grand nombre, ainsi le comité consultatif du secteur financier, fait état d'une baisse tarifaire comprise entre 20 et 41 dont bénéficient tous les assurés depuis 2010 et je crois que nous pouvons nous en féliciter, nous devons cependant améliorer encore davantage le dynamisme de ce marché et la protection des consommateurs est-ce au bénéfice de tous, de nombreux acteurs dans les associations de consommateurs se font régulièrement l'écho de difficultés concrètes rencontrées par nos concitoyens pour substituer le contrat proposé par la banque par un contrat alternatif à travers une délégation d'assurance le dispositif actuel paraît souvent peu lisibles pour les emprunteurs et je suis aussi fermement, fermement convaincus que nous devons continuer à lutter contres les pratiques qui sont de nature à décourager les emprunteurs dans leur démarche le gouvernement soutient donc les mesures qui permettent de rang, le dispositif de résiliation pleinement opérationnel, je pense à la transparence des décisions de refus de substitution pour l'assurance, je pense à la meilleure information des assurés, je pense à l'introduction d'un délai de production de production de l'avenant au contrat de crédit lors d'une substitution d'assurance ou encore au renforcement des sanctions administratives à l'encontre des prêteurs et des assureurs, qui aurait des pratiques dilatoires ainsi conçu le dispositif de résiliation infra-annuelles devra permettent d'accélérer le mouvement engagé en orientant encore les tarifs à la baisse pour le plus grand nombre, cette nouvelle possibilité de résiliation rapprochera aussi l'assurance emprunteur du régime de résiliation infra-annuelles qui s'était ce qui s'est étendu à un certain nombre de contrats de masse comme les assurances auto, les assurances habitation ainsi que les compliments les cette mesure il y a aussi soutenu le pouvoir d'achat, je l'ai dit, c'est peut-être l'objet d'une appréciation un peu divergentes entre monsieur le rapporteur et le gouvernement, mais nous considérons que pour un primo-accédants qui a qui emprunte 250000 euros à 35 ans pour acheter son 1er logement, cette mesure pourrait lui faire économiser sur la durée du prêt d'environ 4000 euros ont au moins 4000 le gouvernement veille enfin tout particulièrement à l'effectivité des réformes menées au bénéfice de nos concitoyens et donc il sera nécessaire de prévoir un bilan de la mise en oeuvre de la résiliation infra-annuelles par exemple un an ou 2 ans après son entrée en vigueur, le gouvernement avait confié au comité consultatif du secteur financier dès l'origine des réformes menées depuis 2010, la tâche de suivre leur mise en oeuvre, je salue l'excellent travail de cette instance, ainsi que les avancées que ce travail a rendu possible. Il y a un 2ème qu'il y a de cette proposition de loi qu'il faut souligner, car il est majeur, vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, il s'agit de permettre aux personnes en situation de risque aggravé de santé du fait d'une maladie ou d'un handicap de pouvoir continuer d'avoir accès à l'assurance emprunteur et donc à la propriété, le Crédit Immobilier de pouvoir être accessible à tous et notamment aux plus fragiles de nos concitoyens, à ce titre, je remercie les parties prenantes de la convention Heras convention signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque de l'assurance de la Mutualité, par les associations de malades et de consommateurs, et qui a pour objet d'élargir l'accès à l'assurance et et à l'emprunt des personnes ayant où il y a eu un problème de santé, leurs travaux ont permis de grandes avancées, les dernières dispositif et dernier dispositif spécifique mis en place depuis 2015 le droit à l'oubli mais également la grille de référence à Heras offrent des possibilités plus large d'accès d'accès à l'assurance des prêts cette grille évolue régulièrement prévoyant la prise en charge par les assureurs et les réassureurs de nouvelles pathologies en fonction des progrès de la médecine et des données de santé disponible ce cadre conventionnel est essentiel pour favoriser l'accès à l'assurance des plus fragiles pour que les candidats à l'emprunt, qui ont été atteints d'un cancer ou d'une autre pathologie ne suffisent pas une double peine avec des refus des exclusions de garantie des surprimes importantes pour raisons de santé, il repose, non sur l'occultation des situations personnelles mais sur l'encadrement des pratiques à l'égard des plus fragiles, c'est pour nous le seul moyen efficace de s'assurer que les assureurs puissent continuer d'assurer les plus fragiles, dans des conditions raisonnables, à l'inverse, modifier un paramètre de ce cadre de manière excessive et injustifiée au regard des données médicales en remettant en cause les conditions de mutualisation d'aléas ne permettrait pas de couvrir davantage les plus fragiles et ce sera dur par un renchérissement massif des tarifs et une suppression de la concurrence puisqu'aucun cas aucun assureur alternatif nourri de de connaissance de ses assurés, nous avons monté depuis 30 ans, toutes majorités confondues, pour un modèle qui repose sur la protection des plus vulnérables, en encadrant les pratiques en intégrant tous les acteurs banque assureur association à une convention de place la collégialité des décisions relatives à l'évolution de la grille de référence à Arras et au dispositif du droit à l'oubli est indispensable, c'est pour nous mêmes conditions pour préserver l'accès le plus large possible crédit des malades et des anciens malades, c'est un modèle qui est copié en Europe car il permet non pas d'ignorer cette situation personnelle vient d'encadrer les pratiques et nous proposons aujourd'hui de renforcer ce régime fondé sur l'association toutes les parties prenantes en traduisant un engagement, un engagement pris par le président de la République, mais un engagement partir de suis partagé par beaucoup sur tous les bancs de l'Assemblée, comme du Sénat, celui de réduire la durée du droit à l'oubli des anciens malade d'un cancer, les malades de l'hépatite C à 5 ans au lieu de 10 et enfin d'augmenter le montant du plafond jusqu'auquel les modalités d'assurance des personnes malades sont encadrés pour mieux les protéger et de le faire en permettant et en prévoyant une méthodologie, vous avez rappelé monsieur le rapporteur, facile, souple, permettant des adaptations, toujours dans le respect du consensus et de l'accord de à ce que j'ai évoqué il y a un instant, vous l'avez compris, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement soutient cette proposition de loi qui amène de la justice qui amène du pouvoir d'achat qui répond à la préoccupation d'un grand nombre de nos concitoyens fragilisés où il en était fragilisé par la maladie et en cela les droits nouveaux que porte ce texte nous paraissent tout à fait essentiel, c'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. Merci monsieur le ministre, je rappelle qu'en application de l'article 42 Alina 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale, le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou accepté par le gouvernement. En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservée, nous passons à la présentation des amendements du gouvernement, avant d'en venir aux explications de vote des groupes Merci monsieur le président, les les amendements du gouvernement d'un objectif qui est soit rédactionnel soit de bon fonctionnement de bonne application du texte, ainsi le 1er amendement propose de supprimer le rapport prévu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour éviter pour éviter la production de rapports différents sur un même sujet, d'autant plus que cette autorité consultée dans le cas des rapports réalisés par le comité consultatif du secteur financier, le second amendement vise à introduire un délai d'entrer en vigueur pour l'article 7 bis, fixé au 1er juin 2022 pour laisser le temps aux professionnels de s'adapter au niveau dispositif introduit par le présent article le 3ème amendement un caractère rédactionnel, le 4ème amendement un caractère rédactionnel et enfin le 5ème amendement propose de préciser la première conditions devaient être respectés pour qu'aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré soit ne soit sollicitée par l'assureur, en précisant que le plafond de 100000 euros s'applique pas rassurés et sur l'encours cumulé des contrats de crédit, c'est le sens monsieur le président, des 5 amendements déposés par le gouvernement. Merci monsieur le ministre, avis de la commission sur le rapporteur.

le délai de 3 mois de l'application sur la fin du questionnaire médical est quelque chose que l'on peut entendre compte tenu de l'importance et les modifications qui d'adaptation pour les assureurs, les bancassureurs, donc c'est un avis favorable de la commission aussi 2ème remarque qui concerne effectivement la demande de rapport de la l'ACPR puisque le sénat avait considéré que ce n'était pas nécessaire, donc on est content de voir que, finalement, on revient à l'idée du Sénat et puis l'autre point, petit détail, et je remercie les services du ministère sur la nouvelle réécriture des 200000 euros,

tant qu'il ne dépasse pas les 200000 euros effectivement et qui ne l'espace passe et l'âge de, de, de 60 ans, donc c'est c'est une précision utile qui évite effectivement pour celles et ceux qui auraient pu abuser du système qu'on avait mis en place, mais qui permet à celles et ceux, effectivement, au cours de la vie de pouvoir se projeter, donc c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, sur l'ensemble de ces amendements. Il monsieur le rapporteur, donc, le vote est donc réservé avec l'ensemble du texte nous passons, explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe. On commence par Florence Béatrix comptable pour le groupe socialiste, écologiste, républicain pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire du 3 février dernier portant sur la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur a été conclusive, je ne peux que m'en réjouir et remercier le rapporteur Daniel Gremillet il y avoir grandement contribué ce texte portait initialement une mesure phare : faciliter la résiliation de l'assurance emprunteur sur le sujet, notre groupe a été à l'offensive depuis de longues années 2014, avec la possibilité de résilier à tout moment à la première année puis 2017 avec l'amendement Bourquin nous saluons donc l'accord trouvé sur le second volet, nous avons collectivement oeuvrer au Sénat, à faire de ce texte, un texte réellement progressiste, j'irai même plus loin, peut-être un texte historique en renforçant le volet santé d'ailleurs, contre l'avis du gouvernement dans un 1er temps donc sur le 1er volet nous avons eu ici un débat sur les modalités de la résiliation majoritairement première lecture notre assemblée avait opté pour une possibilité de résiliation, une fois par an avec une information renforcée et plus clair pour l'emprunteur, l'Assemblée nationale, de son côté a mis l'accent sur la possibilité de résiliation à tout moment, considérant qu'ouvrir davantage la possibilité de résiliation une fluide une fluidité plus importante de ce marché en réalité la concurrence accrue entre assureurs a déjà permis des gains conséquents pour les emprunteurs en moyenne depuis le début des années 2010, monsieur le ministre l'a évoqué, on a constaté une diminution pouvant aller jusqu'à 40 % au bénéfice des emprunteurs et sans baisse de garantie au cours de la commission mixte paritaire, notre souci a été d'encadrer la libéralisation de ce marché afin d'éviter une démutualisation son contrôle et susceptible de nuire à certaines catégories d'emprunteurs, je pense aux plus âgés, ou à ceux ayant des pathologies, donc nous avons veillé à maintenir l'obligation annuelle d'information de l'emprunteur qui reste un autre avis essentiel de même encadre par le prêteur d'une demande de résiliation, il devra justifier intégralement les différents motifs de son refus le se préserver des manoeuvres dilatoires de certains à de certaines banques ou de certains assureurs est essentiel, ces dispositions seront effectives dès 4 mois après la publication de la loi concernant le second volet dans la version initiale de l'Assemblée nationale, pour nous, le compte n'y était pas afin de rendent le crédit plus inclusif aujourd'hui de nombreuses personnes sont exclus de l'accès à l'emprunt et donc de l'accès à la propriété en raison de l'orage, ou de certaines pathologies dont elles ont souffert ou d'être ou dont elles souffrent, nous avons voulu en finir avec cette injustice après la CMP a le travail réalisé au Sénat, il nous faut reconnaître des avancées notables avec notre groupe, nous avions d'abord déposé un amendement pour que le questionnaire de santé soit supprimée pour les prêts inférieurs à 300000 à 500000 euros ça a été finalement 300000 350000 350000 au Sénat et dans le le le compromis le questionnaire de santé supprimer pour les prêts inférieurs à 200000 euros, bien évidemment, nous pouvons regretter ces réductions mais, incontestablement, c'est une avancée et nous sommes persuadés qu'elle en appellera d'autres ultérieurement un autre point important était l'accès à l'emprunt, des personnes qui avaient des pathologies, là encore, nous pouvons exprimer notre satisfaction, le droit à l'oubli, ramené de 10 ans à 5 ans pour les pathologies cancéreuses ou l'hépatite C, c'est vraiment une avancée importante et nous souhaitions néanmoins avancé pour d'autres pathologies, notamment les pathologies chroniques et c'est ce qui sera fait, les partenaires de la convention à Arras, ils travailleront et si les discussions échouent un décret pourra fixer les maladies chroniques auxquels le droit à l'oubli s'appliquera donc en conclusion, au vu des avancées importantes obtenues avec mes collègues sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous voterons avec enthousiasme ce texte et je voudrais terminer en citant Catherine Simonin, administratrice de la Ligue nationale contre concernant ce texte, elle a indiqué une marche de plus a été franchi vers la guérison sociale des personnes ayant eu un cancer et donc je crois que nous pouvons nous féliciter être fiers de ce texte, je vous remercie. la parole est Marie Évrard pour le groupe RDPI pour 6 minutes.

le 26 janvier malgré les profondes modifications apportées par notre vénérable institution à la proposition de loi de la députée Patricia Lemoine j'avais déclaré à cette tribune, faire confiance à la navette parlementaire pour des cadenasser définitivement le marché de l'assurance emprunteur pour le bien des consommateurs, le texte de la commission mixte paritaire du 3 février telle qui nous est proposé atteint pleinement cette autre objectif avec les les sénateurs du groupe RDPI nous sommes satisfaits de l'accord élaboré à l'occasion de cette CMP comme vous avez pu le dire monsieur le rapporteur en commission le 26 janvier dernier : il ne s'agit pas uniquement d'une histoire d'argent, il y va avant tout de l'homme, je partage pleinement votre d'indice je tiens d'ailleurs à saluer votre travail ainsi que celui de la rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin d'aboutir à ce texte équilibré, je vous remercie également madame la présidente de la commission des affaires économiques, pour la qualité des échanges certes les oppositions étaient claires en séance même franche mais toujours courtoise et passer sur de scènes argumentation je n'oublie pas non plus l'engagement et la détermination de Monsieur le Ministre, au-delà des postures politiques trois avancée principale ont su être trouvé pour faire primer l'intérêt de de ses concitoyens, tout d'abord la possibilité de changer à tout moment d'assurance emprunteur va faciliter leur vie, conduire à une baisse des tarifs et rendre du pouvoir d'achat aux Français : nous sommes ainsi au rendez-vous des attentes et de préoccupation de nos concitoyens, le pouvoir d'achat est au coeur des débats pour preuve la 2ème commune de mon département sens a accueilli, jeudi dernier, le 1er ministre à l'occasion du journal de 13 heures de France 2 pour répondre aux questions de 5 Français sur cette thématique, la libération de pouvoir d'achat induite par ce texte, quel que soit son montant ne doit donc pas être négligée, comme vous l'avez indiqué, le 26 janvier cela peut concerner 20 à 25 millions de Français ayant un contrat d'assurance emprunteur actif et sans oublier ceux qui aspirent à devenir propriétaires dans le même temps, la proposition de loi renforce l'information du consommateur sur 6 3 elle alourdit les sanctions pour les établissements bancaires et les assurances qui ne jouent pas le jeu. Elle rend plus transparent, le processus de résiliation de l'assurance emprunteur afin de mettre fin aux mesures dilatoires. Bien connu de tous, l'abaissement du droit à l'oubli de 10 à 5 ans pour tous les malades du cancer et de l'hépatite C, quelle que soit leur âge constitue la 2ème avancée de ce texte, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne des présidentielles de 2017, c'est donc une nouvelle promesse tenue par le président de la République et notre majorité avant la fin du quinquennat cela permettra aux anciens malades du cancer et de l'hépatite C, un accès effectif aux crédits immobiliers, une étape cruciale pour se projeter dans rêve dans l'avenir et se reconstruire sur le plan personnel. Le compromis trouvé concernant la suppression du questionnaire de santé et la 3ème avancée principale du texte, cela concernera les prêts immobiliers jusqu'à 200000 euros pour les personnes de moins de 60 ans, cette question a fait l'objet de nombreux échanges mais au final, nous pouvons nous en réjouir, le texte sur lequel nous allons nous promener prononcé est le fruit d'intenses concertations de bonne volonté transpartisane et du travail en bonne Intelligence de nos de et son impact va être concret dans la vie de nos concitoyens et nous pouvons en être fiers. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Emmanuel Capus pour le groupe, les indépendants pour 5 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'initiative de notre collègue député Patricia Lemoine est une bonne nouvelle pour les Français, je me réjouis de l'accord trouvé en commission mixte paritaire, cette proposition de loi dont nous allons adopter aujourd'hui la version définitive a été soutenu par le gouvernement et enrichi par le Sénat d'apparence technique, elle apporte des solutions très concrètes à des problèmes très concrets avec un objectif clair : rendre l'accès à l'assurance-crédit, à la fois plus simple et plus juste. Les débats que nous avons eues lors de la première lecture l'ont bien montré la réglementation du marché de l'assurance emprunteur repose sur des équilibres délicats entre liberté du consommateur et stabilité des acteurs économiques entre saine concurrence et barrières à l'entrée. Plus fondamentalement, il me semble que cette proposition de loi est un acte fort pour lutter contre les discriminations en raison de la santé, je l'avais dit en première lecture, les discriminations en raison de la santé ne sont tolérés dans un, dans aucun domaine de la société, il n'y a aucune donc aucune raison de les tolérer pour l'assurance-crédit. Pour beaucoup de Français, une maladie passer un cancer vaincu ou même un traitement reste le principal obstacle pour accéder à la propriété. C'est d'autant plus inacceptable que pour des millions de Français, l'achat d'un bien immobilier est un projet engageant qui mobilisent leurs économies et contraint leurs revenus futurs. C'est donc une décision importante et nous devons veiller à ce que personne n'en soit exclu, à raison de son état de santé, il n'est pas juste de renvoyer à leur maladie, passer les axes, les acheteurs qui ont déjà réussi à obtenir un crédit. La mouture finale du texte poursuit cet objectif, le compromis trouvé en CMP me semble équilibré, il a permis de conserver à la fois la mesure essentielle de la proposition de loi initial et les principaux apports du Sénat. C'est pour ma part la ligne que j'avais exactement défendu en première lecture, vous comprendrez donc que je partage tous les points de ce texte, d'une part la possibilité pour les emprunteurs de résilier à tout moment leur contrat d'assurance, cette mesure phare a bien été réintégrées au dispositif législatif et je m'en réjouis, malgré les arguments avancés par nos rapporteurs en première lecture, je reste pour ma part convaincu, il s'agit d'une mesure au service des emprunteurs, c'est-à-dire des consommateurs. Le but n'est pas pour eux de changer sans cesse d'assurance je ne pense pas que les Français vont s'amuser à répéter les démarches administratives en ce sens, en revanche, dès lors qu'ils auront connaissance du une qui leur paraîtra plus intéressante, ils pourront résilier leur contrat sans avoir à prendre date dans plusieurs mois pour changer de contrat d'assurance, telle est le but de cette mesure. Je salue également l'ajout du Sénat concernant la suppression du questionnaire santé pour certains crédits immobiliers. J'avais pour ma part repris un amendement que le Sénat avait adopté lors du dernier budget et qui proposait une solution alternative. Il s'agissait de créer des contrats d'assurance inclusif qui poursuivaient le même objectif, mais qui différaient par la méthode retenue, quoi qu'il en soit, ces 2 mesures permettront de renforcer les droits des emprunteurs de rendre le marché de l'assurance emprunteur plus compétitifs et de faciliter l'accès des Français à la propriété, surtout, elles permettront de lutter contre les discriminations en raison de la santé, vous avez aurez compris le groupe les indépendants votera en faveur de ce texte. Merci, cher collègue, la. Parole est à monsieur Vincent pour les républicains pour 5 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes ici présents pour voter des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple, hein. Et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Le brut, le but 1er était de permettre aux assurés de vouloir résilier à tout moment leur contrat d'assurance emprunteur et d'obtenir un meilleur tarif par le jeu de la concurrence. Actuellement, plus de 88 % des parts de marché sont détenues par les banques qui usent de tous les stratèges il faut répéter pour refuser des demandes de résiliation, bien que la loi le permette le principal stratège utilisé était de refuser au motif que la résiliation non respecté, pas la date d'échéance qui n'existe pas. Bien souvent, ce refus n'était pas acté à l'assuré qu'il se retrouvait donc avec 2 assurances qu'empruntera payer. On comprend alors pourquoi la concurrence est vite découragé sur le sujet. Et pourquoi les banques ont maintenu un niveau de cotisations élevées par rapport au sinistre niveau de sinistres à primes, comme on dit dans notre jargon qui est de 34 % et donc très rentable. Alors que le texte de l'Assemblée nationale visait à permettre à la résiliation à tout moment à informer d'assurer du refus de résiliation dans un délai court, a fixé un délai de 10 jours à la banque pour éviter de nouvelles avenant du prêt avec délégation d'assurance, nous pouvons nous féliciter de ces avancées et approuvons les articles en ce sens, qui vont donc libéraliser ses assurances et garantir un meilleur tarif aux assurés. La première partie du texte avait le mérite de répondre à un accès plus simple et plus transparent à l'assurance emprunteur, mais pas à un accès plus juste, comme le veut le titre. Il a fallu attendent le texte du Sénat et de son rapporteur Daniel Gremillet pour y répondre en 2ème partie. Vous allez sûrement être surpris par ma position, en effet, je vous rappelle qu'avant d'être sénateur, je suis agent d'assurance et qu'à plusieurs reprises, j'ai vécu des situations difficiles, comment expliquer à une personne, quel que soit son âge, qui a été atteint d'un cancer, qui est en rémission depuis plus de 5 ans, qui se rend à chaque contrôle semestriel avec l'angoisse de la rechute qui reçoit, après quelques jours, des bons examens qui, encouragé par ses médecins pour prendre pour reprendre foi en l'avenir, envisage d'avoir des projets personnels et professionnels, comment expliquer à cette personne qui ne pourra obtenir son prêt professionnel parce que le questionnaire médical mentionne sa pathologie, même si elle est très ancienne et que qu'un assureur, acceptera de prendre de risque. Imaginez leur désespoir et leur impossibilité à penser à autre chose que leur maladie pendant toute leur vie, ils ne peuvent devenir propriétaires dans leur vie privée, et ils ne peuvent construire une vie professionnelle. Ces situations sont humainement insupportable pour l'assurer, le banquier, l'assureur, je tiens à le dire. Ce sont les apports du Sénat et de notre rapporteur, nous n'aurions pas régler le problème, nous aurions continué de notifier des refus aux personnes atteintes de maladies pour l'acquisition de la résidence principale et pour ceux qui ont été malades depuis plus de 5 ans. C'est une avancée considérable pour les assurés, bien plus importante que de résilier à tout bon. Monsieur le Ministre, je n'ai pas compris la position du gouvernement sur votre refus de l'article 7 du texte qui impose aux assureurs de souscrire des contrats sans questionnaire médical à toute personne qui veulent emprunter pour leur résidence principale, je n'ai pas compris votre refus du droit à l'oubli des pathologies cancéreuses au-delà de 5 ans. Par ces articles nous répondions à une vraie attente des Français. Vous avez prétexté que le but recherché de diminuer le tarif en simplifiant l'accès à la résignation. Et qu'en intégrant cet article, les assureurs, les assurés à les payer plus cher vos arguments ne tiennent pas. Vous regrettez juste je pense, de ne pas avoir eu l'idée avant les les sénateurs. Pourtant, vous le savez, il fallait que les textes de loi impose cette obligation aux assureurs pour que les conditions et pour imposer soient les mêmes. Et pour qu'il le calcule un tarif par rapport à une population plutôt qu'à une personne, et quant à la hausse du tarif, nous pouvons avoir des doutes, compte tenu de la marge bénéficiaire existante, à nouveau, au risque de me répéter. Je félicite le rapporteur Daniel Gremillet, et le Sénat de cette avancée et de nord pas céder sur ce sujet, au risque de rendent la CMP non conclusive. père plane, le Parlement a pleinement exercer son rôle et l'objectif visé de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur a été pleinement rempli avec le groupe des Républicains nous voterons donc les conclusions de cette commission mixte. Merci,

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, nous nous félicitons avec le groupe Écologie Solidarité territoire que la commission mixte paritaire et réussi à trouver un accord. Sur cette proposition de loi sur l'assurance emprunteur un sujet important pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, pour ceux qui s'engagent dans un prêt bancaire. Nous soutenions la disposition phare du texte initial, article 1er prévoyant d'ouvrir la possibilité de résilier sans frais, il y a tout moment les contrats d'assurances emprunteurs pour des crédits immobiliers et non plus seulement au cours de la première année ou à l'anniversaire du contrat, cette mesure a fort heureusement été maintenue dans le texte final, la majorité sénatoriale ayant privilégié le statu quo de la résiliation annuel, le risque de la démutualisation n'est pas avéré au final, seuls les assureurs ou courtiers qui excluait les personnes en mauvaise santé devront désormais intégrer le coût de ce risque dans leurs tarifs, les banques françaises ne verront pas leurs tarifs augmenter brutalement car elles intègrent déjà les emprunteurs malades et mutualistes fortement les risques, il s'agit là d'une mesure de bon sens, attendu par les Français, qui devrait porter ses fruits rapidement, nous l'espérons, nous saluons également les dispositions du texte pour rendre l'assurance emprunteur plus accessible aux personnes les plus fragiles et à celles qui présentent un risque aggravé de santé en ce sens, réduire de 10 à 5 ans la durée de droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses et étendre ce droit à l'oubli à l'hépatite C sont des mesures justes et attendue. Si nous regrettons qu'il n'ait pas été élargi également aux maladies chroniques et au VIH, nous faisons confiance aux membres de la convention qui désormais doivent se saisir de cette question pour que les négociations aboutissent à un accord, autre point majeur du texte, la suppression du questionnaire de santé pour les prêts d'un montant inférieur à 200000 euros par personne et pour les personnes de moins de 60 ans, ce qui constitue là aussi une belle avancée, de justice et de solidarité, même si sur ce point, le Sénat avait été encore plus ambitieux quant au plafond de quotité et d'âge, la mesure adoptée représente quand même une avancée notable, ce questionnaire dans lequel il est demandé aux clients de dresser l'historique de leur antécédents visite médicaux permettait aux banques de mettre en place une tarification au risque. Généralement très défavorable aux personnes atteintes de maladies longues ou chronique qui se retrouvaient même parfois totalement exclues du marché de l'assurance emprunteur. Comme le soulignait monsieur le rapporteur, les assureurs n'ont pas besoin de 10 pour disposer d'autant d'informations pour tarifer le risque présenté par un assuré au final si nous aurions préféré aller plus loin sur le droit à l'oubli et le questionnaire de santé ou encore sur les questions de transparence, nous voterons pour ce texte qui aurait été réintégré sa mesure phare, la résiliation de l'assurance emprunteur à tout moment et qui s'est enrichi des apports pertinent porté par notre rapporteur après plusieurs lois successives, la libéralisation du marché de l'assurance emprunteur immobilier n'était toujours pas au rendez-vous, nous espérons que ce texte permettra réellement de débloquer la situation et qu'il entraînera un transfert de revenus non négligeable des banques vers les emprunteurs grâce à une véritable mise en concurrence et participera ainsi à la lutte contre contre les rentes bancaire. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Allez,

monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Nous aussi nous nous félicitons de l'Accord trouvé en CMP, qui va rééquilibrer la relation entre les banques, assureurs et l'emprunteur nous remercions sincèrement notre rapporteur pour ces travaux et, surtout, nous pensons que c'est une bonne chose pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui pourront est maintenant à tout moment leur assurance emprunteur, comme nous l'avions proposé et si j'étais un peu taquin, je dirais à la majorité sénatoriale, écoutez un peu plus le côté gauche de l'hémicycle, on aurait trouvé un accord à un peu plus rapide en CMP, mais c'est évidemment. Un peu taquin, par conséquent, nous saluons cette avancée qui permettra aux ménages éloignée des pratiques de l'assurance de bénéficier de meilleurs tarifs et de sortir de l'emprise des établissements bancaires par ce texte, nous admettons enfin que les pratiques dilatoires des banques sont inhérentes à leur situation, ultra-majoritaire les Blank définit les prix, il n'y a pas de fluidité du marché, car les gens se ne dispose pas de l'information nécessaire ne connaissent pas les conditions de garantie et les règles du marché et, enfin, les banques s'arrogent les meilleurs contrats et laisse gérer le risque aux assureurs alternatif non la concurrence pure et parfaite n'était pas une réalité si nous devons choisir de consacrer un droit de résiliation à tout moment, il n'en demeure en pas moins qu'il faut accroître l'information des consommateurs grâce aux propositions notamment du rapporteur ici au Sénat, nombre de nos concitoyens subissent des discriminations en raison de leur état de santé et se voient appliquer surprime et exclusions de garanties disproportionnée, c'est absolument intolérable à ce titre, nous saluons l'avancée réelle du raccourcissement du droit à l'oubli de 10 à 5 ans pour les cancers et l'hépatite C, que nous avons voté ici-même à l'unanimité l'administratrice de la Ligue nationale contre le cancer, Catherine Simon a a eu même des mots très justes, en affirmant que la guérison médicale se traduira un peu plus par une guérison sociale la suppression du questionnaire de santé s'inscrit là aussi dans la même voie, réduire les discriminations sous une forme de condamnation à perpétuité social lorsqu'on est, où nous avons été malade, je sais que les associations de malades et nos concitoyens les plus atteints, les plus vulnérables pâtissent du comportement des Boks des banques, pardonnez-moi, à leur égard, la peur doit changer de camp, pour autant, il nous faudra être attentif sur cette mesure que nous avons voté collectivement et s'assurer qu'elle aura bien et que le roi bien pardonnez-moi les effets attendus parce qu'il y a quelques risques d'effets de bord je m'explique : la suppression du questionnaire pourrait engendrer une hausse générale du coût de l'assurance pour tous nos concitoyens, alors aurait beau jeu en expliquant qu'elles répartissent les risques d'augmenter les tarifs, il faudra que nous y soyons vigilants, la suppression 2ème du questionnaire de santé pourrait également détourné la volonté d'assurer des banques à des profils qui, a priori, représente le moins de risques de santé, les jeunes, les cadres, l'ancienneté sur un poste laissant toujours davantage les assureurs alternatif ce préoccuper des éloigné de l'assurance et donc de l'accès au crédit immobilier, une dernière chose qui nous tient à coeur à nos groupes, c'est évidemment que nous allons supprimer le questionnaire de santé, mais ne rêvons pas : les banques disposent de nos données de paiement, là aussi, il faudra être extrêmement attentifs, car c'est une mine d'or pour un certain nombre de banques qui peuvent savoir combien de fois nous allons à la pharmacie, combien de fois nous allons au médecin à l'hôpital ou pour aller au tabac ou tant d'autres choses, il faudra donc être extrêmement vigilant et là, le suivi de la loi sera extrêmement important enfin pour générer de l'inclusion, il faut s'évertuer à rendre accessible assurance par l'obligation d'intégrer les profils dits à risques, comme nous le proposions il faut donc que chaque emprunteur dont la demande de crédit a été acceptée, se voit proposer une assurance emprunteur aux garanties minimales sans surcoût ni surprime avec l'ensemble de ces questions, nous sommes d'accord et réjoui de voter cette CMP, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur permet d'illustrer tout l'intérêt d'un bicamérisme apaisé et constructif, en effet, et comme cela vient d'être rappelé le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, compromis qui n'était pas écrit d'avance, je crois pouvoir dire que nos 2 chambres ont chacune fait un pas l'une vers l'autre, donc dans les dispositifs qui nous sont proposées, ce rapprochement a été possible, car sur le fond, les objectifs de cette réforme de l'assurance emprunteur immobilier étaient les mêmes pour les députés et pour les sénateurs, à savoir garantir le meilleur niveau de protection de l'emprunteur au coût le plus juste, simplifier les processus d'acquisition et de résiliation d'assurances en garantissant la transparence des décisions. Améliorer l'information du consommateur tout au long de son contrat d'assurance avec mes collègues du groupe Union centriste et en particulier Sylvie Vermeillet ces axes constituait déjà notre boussole lors de la première lecture de la proposition de loi, nous sommes en effet convaincus que ces objectifs sont plus important encore que les mesures précises qui étaient proposé ainsi le texte finalement réécrit présente de grandes avancées en matière de droit de la consommation en faveur de l'ensemble des emprunteurs, à ce titre, il constitue l'aboutissement de toutes les évolutions législatives depuis 2011 après les lois Lagarde et Hamon après l'amendement Bourquin nous allons adopter aujourd'hui la dernière brique d'un ensemble législatif cohérent et qui est toujours allé dans le même, la même direction. Ne tombons donc pas dans le piège d'opposer, députés et sénateurs ou de créer de fausses polémiques nos 2 chambres ont toujours fait le même choix, améliorer le droit des consommateurs. Salon ainsi l'équilibre trouvé qui permettra désormais de résilier à tout moment les contrats d'assurance emprunteur comme voté par l'Assemblée nationale, mais avec des obligations d'information des assurés sur leurs droits à résiliation comme adopté par le Sénat. Le texte valide aussi la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieur à 200000 euros, comme proposé par la commission des affaires économiques du Sénat, enfin il réduit de 10 à 5 ans le délai de droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses et l'hépatite C, telle que souhaitée par le Sénat. Ces 3 mesures phares répondent de manière très claire aux difficultés existant aujourd'hui pour les emprunteurs, celles-ci sont en effet le manque de transparence des dispositifs existants et des décisions des banques, la faiblesse de l'information du consommateur et les freins dans l'accompagnement des publics les plus fragiles sur ce dernier point, le Sénat a vraiment fait oeuvre utile et Ada et d'avant-garde personne avant l'examen de cette PPL n'aurait imaginé que le texte final soit si ambitieux sur le droit à l'oubli et pour les personnes les plus pénalisé par les pratiques actuelles. La suppression du questionnaire médical est une belle porte ouverte, c'est une vraie mesure d'accompagnement social, aujourd'hui, à l'origine d'inégalités fortes entre les consommateurs, naturellement, il faudra revenir sur les seuils fixés en matière de montant et concernant l'âge dès que nous aurons les premières analyses sur les conséquences de ce texte, nous comptons sur ce point sur les pouvoirs réglementaires à qui nous avons fixé un objectif d'adaptation, de manière à réussir cette réforme sur ce point précis, comme sur le reste du compromis du compromis j'aimerais saluer le travail et l'engagement de notre rapporteur Daniel Gremillet, il n'a pas ménagé sa peine pour aboutir à un texte commun et surtout défendent la singularité, les apports du Sénat, en conséquence, vous l'aurez compris le groupe Union centriste votera en faveur des conclusions de cette CMP, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est au président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous aurions après plusieurs mois de débats passionnés à l'examen des conclusions de cette proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple, plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, hé bien à ce sujet au nom de mon groupe, a salué l'immense travail réalisé par les 2 rapporteurs de notre collègue sénateur Daniel Gagnier et la députée Patricia Lemoine cette volonté commune d'avancer. A permis de réunir une commission mixte paritaire dans un adversaire constructive aussi j'ai des investissements et tout à fait louable dans le marché de l'assurance emprunteur concerne des millions de Français sur tout le territoire, ce que faisait assurance ne soit jamais ne faut pas juridiquement obligatoire, elle est très courant lors de l'octroi d'un prêt immobilier, nous dirons donc l'impact significatif de ce texte dans la vie quotidienne de bon nombre de nos concitoyens,

impliquant souvent ou d'avoir recours à l'abri, si les marchés du recours à l'emprunt s'ajoutent traditionnellement à d'autres démarches de nature administrative, au cours desquels nous faisons face à d'innombrables demandes de pièces justificatives des difficultés à contacter un interlocuteur des mauvaises informations etc pour lui en effet le sentiment d'un parcours du combattant, notamment pour les foyers modestes la présente proposition de loi rejeté ainsi à nos yeux une importance capitale concernant le renforcement des prérogatives des emprunteurs face aux assureurs, force est de constater que l'accord trouvé un 2ème bébé, répond positivement à cet objectif pour rappel lors du 1er examen dans cet hémicycle, notre groupe s'étaient abstenus en raison du désaccord avec la majorité sénatoriale sur la rédaction de l'article 1er substance de la proposition de loi, le retour à la version initiale du texte, je suis oui suite à la plaît avec une possibilité de résiliation à tout moment des contrats d'assurance emprunteur, assorti d'une obligation. Pour l'assureur d'informer chaque année l'assuré de son droit nous satisfait, cela contribue non seulement à accorder plus de liberté aux assurés, mais cela va également dans le salle de l'amélioration de l'accès au droit, le rétablissement de l'article 3 bis prévoyant la mention obligatoire du coût de l'assurance, sur une durée de 8 ans constitue une sécurité supplémentaire pour les assurés et leurs ressources en août, nous accueillons positivement la rapidité avec laquelle les mesures contenues dans le titre 1er de cette proposition de loi entre en vigueur, grâce à l'article 6 sur le volet médical, la réduction de 10 à 5 ans après la fin du protocole thérapeutique de la durée du droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses et ça, si on ne ce droit à d'autres pathologies comme l'hépatite C, est un progrès incontestable, c'est une très belle Exposition et une protection essentielle en direction des emprunteurs qui ont été affectés par le passé par certaines maladies, d'autre part, le président texte prévoit un plafond de 200000 euros

de ces 200000 euros 193204 euros en 2021 et le terrain toutefois nous serions la nuance apportée avec la possibilité pour le pouvoir, der de faire évoluer à la hausse après étude du comité consultatif du secteur financier et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à propos d'évaluation, l'obligation de la réalisation d'un rapport 2 hommes après la promulgation de la présente loi nous permettra d'identifier les outils les plus efficaces au vu il y a l'objectif originel, sommes nous vous l'avez compris notre gros porteurs regard favorable ah oui à cette assure équilibré de la proposition de loi réformant le marché de l'assurance emprunteur et donc nous voterons pour ce texte. Merci, cher collègue. Je donne la parole à la présidente de la commission. dans son intervention ne correspondent pas tout à fait aux chiffres qui nous ont été données par les services de Bercy, ce que vous annoncez est annoncé dans l'UFC que choisir, mais nous, nous avions des informations des services de de vos services qui disent que l'économie substantielle serait à peu près 2300 euros par ménage, c'est beaucoup, on y fait attention mais ça ne fait pas les 550 millions que vous annoncez en tout cas le Sénat sera attentive, vous l'avez compris à haut risque de démutualisation de cet article 1 et les rapports de suivi seront donc les bien venus, je voulais vous dire mais comme mon mon collègue Fabien gage je serais un peu taquine que vous vous félicitez de cette proposition de loi que nous allons à priori voté à l'unanimité, mais je voudrais quand même rajouter qu'il a fallu combattre pied à pied et rendre hommage au travail de Daniel Gremillet, pour que nous y arrivons, mais face à Seguin a dit cela parfaitement tout à l'heure, je ne vais pas en dire davantage, ensuite je voulais vous dire monsieur le ministre, que vous avez beaucoup parlé de la convention à grâce à juste titre d'ailleurs, je voulais vous dire que quand même dans les auditions 100 % des associations 100 % des associations nous a indiqué que la convention ne répondaient pas à leurs questions et à leurs besoins et donc ce procès de propositions de loi que nous nous apprêtons à voter va leur donner un sérieux coup de main dans la négociation et, dans le cadre de cette convention, à Arras, donc je suis, je pense que nous allons cet après-midi, faire oeuvre utile pour une 2ème fois dans l'après-midi peut-être voté à l'unanimité du Sénat une 2ème CNP et donc je suis vraiment très reconnaissante au travail de Daniel Gremillet au travail des services du Sénat Laurent qui est bien sûr la comme administrateur mais je voudrais aussi avoir une pensée pour pour notre collègue Martial Bourquin, qui a initié cette démarche, il y a quelques années et qui voit qui se voit se se terminer aujourd'hui voilà donc merci à tous, merci de votre soutien merci à l'ensemble des groupes du soutien et merci, cher Daniel. Merci madame la présidente. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission sur l'ensemble du texte, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Voici les résultats des scrutins 106 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs au politique et notifié à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 343 pour l'adoption 343 contre 0, le Sénat a adopté. Chers collègues, je vais suspend la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Monsieur le président, madame la rapporteure chers Anne-Catherine voici mesdames, ces messieurs les sénateurs, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le léger retard avec plus de 17 millions d'hectares en métropole et 8,7 millions d'hectares en Outre-mer, la forêt française constitue un atout stratégique pour la France en tant qu'ingénieurs agronomes et forestiers ma vision pour la forêt est très clair nous devons préserver ce qui fait la richesse plurielle de nos forêts, notre forêt possède en effet une triple fonction, une fonction environnementale avec une grande capacité de stockage de carbone et des atouts indéniables pour préserver la biodiversité une fonction de ressources naturelles ensuite au service par exemple de la construction bois de l'utilisation de ce si beau matériau qui est le bois et vous le savez mieux que quiconque le bois constitue un matériau de choix dans le cadre de la lutte contre le changement climatique grâce à ses capacités à stocker du carbone et enfin une fonction sociétale, très importante pour l'ensemble de nos concitoyens et aucune de ces 3 fonctions environnementales économique, c'est-à-dire de ressources naturelles, mais également sociétale ne doit être oublié, c'est bien cette richesse plurielle qui est sculpté nos forêts et qui a sculpté nos politiques forestière et de la filière bois alors dans chaque territoire l'importance de chacune de ces 3 composantes peut varier mais nos outils de gestion doivent permettent de faire vivre cet équilibre et de s'adapter à la réalité de chacune de nos forêts, la gestion durable des forêts sur ces 3 volets environnementaux, économiques et sociaux est à ce titre essentiel et le code forestier dont nous allons discuter défini ainsi des conditions rigoureuses de reconnaissance et lui, exercice de l'ensemble de ses activités cultiver notre forêt cultiver notre forêt et et nécessite d'avoir une bonne gestion et donc, par exemple, des actions de renouvellement, ce n'est pas une soirée sous cloche, c'est ce travail important de protection et de culture que mène au quotidien les exploitants forestiers avec passion et envie de transmettre un Patrimoine de qualité aux générations futures, alors pour relever ce défi d'une gestion multi-factorielles, l'État se mobilise et investit massivement en faveur de la filière forêt, Bois, notamment au travers du plan de relance, nous avons consacré plus de 150 millions d'euros à cet enjeu du renouvellement forestiers pour remplacer des peuplements qui parfois dépérissent, du fait du changement climatique, à ce jour plus de 90 millions d'euros sont d'ores et déjà engagés pour des projets concrets dans les différentes forêts qu'elle soit domanial communal ou privé et si ces résultats sont satisfaisants, je compte sur la mine, la mobilisation de toutes et tous pour maintenir cette dynamique, car en effet, le président de la République a annoncé il y a déjà plusieurs mois que de le cadre de ce grand projet, France 2030, c'est plus de 600 millions d'euros supplémentaires qui seront déployés sur les prochaines années, au bénéfice de nos massifs forestiers et de notre filière bois je crois que c'est extrêmement important et je crois aussi que nous pouvons dire que jamais nous n'avons autant investi pour nos forêts avec, au final, c'est 800 millions d'euros d'investissement qui sont d'ores et déjà engagés ou en cours d'engagement alors pour déployer tout cela il nous faut le faire dans le dialogue dans le dialogue entre tous les acteurs, cette véritable dynamique faire filières qui est un enjeu incroyablement important pour cette filière forêt, Bois afin d'avancer ensemble dans la gestion des enjeux et répondre à des questions opérationnelles en dépassant les multiples rapports qui ont été faits sur la forêt pardon des conditions de ce dialogue constructif, la véritable dynamique au sein de cette filière bois sont au coeur de notre action ces derniers mois et je voudrais à ce titre, citer 2 exemples d'abord cet accord de filières à destination du chêne, que nous avons signé ce matin avec l'ensemble des parties prenantes de la filière, vous savez, dans une situation combien compliqué du fait des exportations, pardon, de plus en plus massive de nos chaînes vers d'autres pays, notamment en Asie, cet accord de filières est en tous points, je crois, exemplaire parce qu'il montre la mobilisation de l'ensemble de la filière de l'amont à l'aval pour faire face à un défi qui est devant nous et qui est un déficit d'ailleurs à la fois environnemental et de souveraineté mais également 2ème Exemple cette belle dynamique que nous avons lancé et vous y avez participé, c'est-à-dire ces assises de la forêt du bois qui sont en cours, des assises que nous pilotes ont, avec mes collègues Bérangère Abba, Agnès Pannier-Runacher, Emmanuelle Wargon, et qui dans l'ensemble de leurs travaux, confirmé la qualité des contributions, la qualité des discussions et surtout la vision d'actions concrètes concrètes à mettre en oeuvre pour faire avancer la filière forêt la filière bois, ces assises constitue un espace permettant d'associer les territoires pour nourrir la vision la plus large possible de cette forêt française et de la filière bois d'aujourd'hui et de demain et nous allons clore cet exercice dans les prochains jours dans les prochaines semaines et je voudrais, à titre personnel, remercier très spécifiquement Madame la rapporteure pour son engagement dans ces assises je sais toute la passion et l'énergie de Madame la rapporteure sur ces questions de forêt et du bois et en tant que président d'une des thématiques de ces assises, je voudrais souligner à quel point elle joue un rôle déterminant dans la réussite de ces travaux et je voulais vous en remercier depuis cette estrade et là encore, aujourd'hui madame la rapporteure, vous montrez votre engagement et votre volonté d'agir pour nos forêts puisque l'une des difficultés, pas la seule, mais l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et la question du morcellement de la forêt française et à ce titre-la proposition de loi que vous étudiez aujourd'hui est importante au regard du rôle que jouent et doivent jouer encore plus demain qu'aujourd'hui, face à ces enjeux, les experts forestiers, des organisations de producteurs et les gestionnaires forestiers professionnels, cette proposition de loi doit permettre à ces acteurs de mener efficacement leurs actions d'information à destination des propriétaires forestiers privés et contribuer ainsi à la gestion durable forestière et cette proposition de loi donnera un accès illimité à ses secteurs forestiers reconnue d'intérêt général aux données utiles du cadastre la loi d'avenir pour l'agriculture, de l'alimentation et la forêt de 2014 et son décret d'application de 2016 prix après l'avis favorable de la CNIL, on termine d'expérimenter cette accès pendant 3 années pour ces acteurs forestiers mais le retour de cette expérimentation devait être fait valider par la loi et le fait que cette proposition de loi le permet, est extrêmement positif, la matrice cadastrale est en effet le seul instrument qui permettent d'identifier les propriétaires des parcelles forestières, or la forêt française est extrêmement morcelé, morcelé, plus de 3,5 millions de propriétaires forestiers et le nombre de propriétaires peut-être important sur une surface très réduite, ce dispositif expérimental a permis d'initier des actions dans des zones forestières non géré depuis des décennies, permettant ainsi d'identifier, d'informer, puis de mobiliser des propriétaires forestiers au service de la gestion durable de nos forêts, alors que ne ne nous ne les connaissions pas, et parfois même eux-mêmes n'étaient pas forcément informés qu'il était : les propriétaires de tels espaces et et morceaux de parcelles forestières alors la pérennisation de l'accès telle qu'expérimentée fait donc pleinement sens pour le gouvernement, c'est pourquoi je vous propose d'adopter cette présente proposition de loi en réitérant mes remerciements spécifiquement Madame la rapporteure c'est beaucoup une nouvelle fois impliqué sur ce sujet, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, la parole est donc Anne-Catherine Loisier, rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui la proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales présenté par le député Nicolas Turquois et adopté en janvier 2021, à l'Assemblée nationale, elle a pu être inscrite in-extremis alors à l'ordre du jour des travaux du Sénat alors que l'actualité, vous l'avez dit, monsieur le Ministre de la filière bois, plaide aujourd'hui pour une meilleure gestion durable de cette ressource naturelle, cette proposition de loi dont le titre n'est pas très approprié puisqu'elle concerne en fait l'ensemble des gestionnaires agréé et pas uniquement les experts forestiers reprend le dispositif d'un amendement sénatorial transpartisan adoptées dans la loi d'avenir pour l'agriculture à la forêt de 2014, il prévoyait à l'époque une expérimentation triennal simplifiant l'accès aux données cadastrales pour les experts forestiers, les organisations de producteurs, les gestionnaires forestiers professionnels, l'objectif était déjà de favoriser la gestion regrouper des parcelles et de lutter, lutter ainsi contre les conséquences du morcellement de la propriété forestière privée, à savoir l'absence de gestion durable le plan cadastral et bien évidemment déjà ouvert au public mais les données littéral du cadastre, dont l'identité et les coordonnées des propriétaires ne le sont pas, au nom de la protection de la vie privée, la mesure proposée en dérogeant au principe facilite l'identification des petits propriétaires de parcelles non gérés par les gestionnaires afin de les informer des modalités d'accompagnement existantes, ces petits propriétaires, vous l'avez dit, monsieur le Ministre méconnaissent souvent en effet, même l'existence de ces parcelles et a fortiori les possibilités de gestion durable l'enjeu autour de la gestion de ces petites parcelles forestières et majeur, la forêt française est au 3 quarts privé 12 millions d'hectares en métropole pour 3 millions et demi de propriétaires et seulement 3 millions d'hectares disposant d'un PSG si l'on décompte les quelques millions d'hectares gérée sous code de bonnes pratiques sylvicoles, c'est dire l'importance de ces dormante ne bénéficiant pas d'une gestion durable suivi ce sont des parcelles timbre-poste ou encore des bandes de forêts, de quelques dizaines de mètres de large et parfois plusieurs kilomètres de long, issus de découpage et de succession, beaucoup d'efforts sont menées depuis des années par les pouvoirs publics, le Centre national de la propriété forestière, les régions, les départements, au travers de stratégies locales de développement forestier pour lutter contre ce morcellement synonyme de non gestion les tensions grandissantes d'approvisionnement en matières premières bois amène aujourd'hui les pouvoirs publics a cherché à mobiliser plus et à mobiliser mieux la ressource les ressources existantes sur l'ensemble du territoire ainsi la valorisation de la forêt et les moyens de garantir son approvisionnement font depuis octobre, l'objet d'intenses discussions dans le cadre de ces assises de la forêt du poids que vous avez initiée, monsieur le Ministre, avec 3 de vos collègues, les réflexions ont largement porté sur une meilleure valorisation de 6 millions d'hectares de forêts puits de carbone et de ressources qu'il est devenu aujourd'hui essentiel de mettre au service des enjeux sociétaux l'article unique de la proposition de loi que nous examinons est strictement le même que l'article voté dans le projet de loi ASAP moyennant tout de même 2 ajouts par l'Assemblée nationale en première lecture, auquel le Sénat est favorable, à savoir en tout cas, la commission des affaires économiques et favorable, à savoir un avis de la CNIL et une date butoir de 6 mois pour prendre le décret, je voudrais en quelques mots : revenir sur quelques éléments de cadrage de cette proposition doit qui peuvent prêter à débat, à savoir le périmètre même de la dérogation qui se justifie au regard des objectifs d'intérêt général et les conditions énumérées par la CNIL concernant le périmètre de la dérogation en permettant la mise en gestion durable de parcelles forestières jusque-là abandonner cette proposition de loi est une réponse aux enjeux de lutte contre les émissions de gaz à effet, effet de serre d'adaptation au changement climatique, tout autant que de valorisation d'un matériau renouvelable, nous connaissons tous, chers collègues, des risques croissants d'incendies dans les forêts non gérer nos forêts seront d'autant plus résilientes qu'elles seront gérées et adapter progressivement aux changements climatiques, nous entendons les besoins de notre industrie pour approvisionner en matériaux durables, les besoins des filières construction, bâtiment emballages ameublement, nous avons largement débattu dans la loi climat et résilience de la nécessaire optimisation des fonctions de puits de carbone et de séquestration des écosystèmes forestiers, l'objectif est, je le rappelle, de passer de 2 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui séquestrés chaque année à 20 millions en 2050, soit une multiplication par 10 en à peine 30 ans en ce sens les plan France relance et France 2030 investissent aujourd'hui massivement dans la modernisation de la filière pour accompagner cet allongement de la durée de vie des produits afin de séquestrer le carbone plus longtemps en promouvant la mixité des matériaux dans la construction, la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, l'air va va entrer en vigueur au 1er janvier permet de substituer permettra surtout de substituer davantage de matériaux, bois renouvelable au traditionnel matériaux plus émissifs ces dernières années, avant les dépérissements massifs liés au réchauffement climatique, la récolte annuelle n'équivalait pas à l'grâce à l'accroissement naturel annuel des forêts, c'est dire que la forêt française est loin d'être surexploités en gérant plus et mieux nos forêts nous préserverons un capital forestier devenu plus vulnérable du fait des fortes chaleurs des déficits hydriques et des attaques d'insectes répéter notre collègue Daniel Gremillet rappelait fort à propos, en commission, combien l'accès des chambres d'agriculture aux données du cadastre, avaient pu être utile après la tempête, tempête de 99 pour identifier les parcelles touchées extraire les chablis et procéder au reboisement, c'est bien parce qu'elle contribue à ces objectifs publics prioritaires que la simplification de l'accès au cadastre pour les gestionnaires agréé est jugée conforme au droit par la CNIL dans ces 2 avis de 2014 et 2015, cette dernière précise bien que seuls des organisations relevant d'une mission d'intérêt général tels que celles agréées par une autorité administrative ordinale retenus dans le cadre de cette loi serait légitimement habilité à accéder à ces données, d'autant que ses prérogatives élargies vont désormais, notamment depuis la mise en place du RGPD en 2018 aller de Pair avec une responsabilité élargie en ce sens, la commission des affaires économiques souhaiteraient un engagement de votre part, monsieur le ministre pour que votre administration accompagne la filière dans l'élaboration d'un code de bonnes pratiques favorisant l'appropriation par les gestionnaires forestiers des règles fixées dans la loi dans le décret et par la CNIL, cette proposition figurait d'ailleurs déjà dans un rapport du CGER en 2019, de bonne pratique pourrait ainsi opportunément clarifier la distinction essentielle entre l'information à diffuser et le démarchage commercial abusif elle rappellera les sanctions administratives voire pénales en cas d'utilisation des données cadastrales à d'autres fins que la gestion durable et elle définirait enfin des modalités de suivi et d'évaluation des impacts de la mesure moyennant ces précautions d'usage qui nous semble nécessaire à la bonne application et la bonne mise en oeuvre de la loi, la commission des affaires économiques, s'est prononcée favorablement pour cette proposition de loi, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame à monsieur Christian Redon Arazi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, je me félicite de voir cette proposition de loi qui vise à pérenniser une habilitation votée dans la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 un truc donc à notre hors du jour introduite sous le quinquennat précédent elle permettait aux experts forestiers, l'accès aux données cadastrales afin de mener à bien leur mission, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de solidifier dans notre droit, cette expérimentation qui, depuis, pardon a été unanimement reconnues comme positives, tandis qu'en parallèle, les experts forestiers ont demandé la prolongation, leur demande est légitime ces derniers participent à la protection et à la mise en valeur des bois et des forêts, ainsi qu'au reboisement, dans le cadre une gestion durable de nos forêts, en effet, ils font face au très fort morcellement de la forêt privée française caractérisée par un nombre très important de propriétaires trop souvent peu, voire mal identifié notre pays doté de la 4ème surfaces forestières d'Europe compte près de 4 millions de propriétaires qui se partagent 76 % de la surface forestière privée. Ce morcellement est un frein à la fois à la mobilisation de la matière première en France, dans un contexte, du moment que l'on connaît, concernant la demande, mais également au bon entretien de nos forêts, les rampes de fait plus compliqué l'exercice des missions des experts forestiers qui doivent avoir accès à certaines données pour les mener à bien. Je salue donc le choix du rapporteur et du gouvernement de s'en tenir à la rédaction de 2014, c'est-à-dire donner aux experts forestiers l'accès sans limitation du nombre des demandes aux données cadastrales des propriétés font forestière dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leur mission d'information, de fait, les garde-fous alors mises en place ont été conservés, le rôle du maire est ainsi préserver celui-ci devant être notifiés lorsqu'il ne demande à l'UE dans sa commune, les données quant à elle, ne pouvant par la suite être cédées à des tiers en nous tenant à la rédaction d'origine nous restons conforme à l'avis rendu par la CNIL, lors du vote dans la loi pour l'avenir de l'agriculture, ce texte donc permet, par le biais des experts forestiers et du maintien de ce droit d'apporter une aide aux petits propriétaires face au morcellement de nos forêts sans pour autant tomber dans une logique de seule rentabilité que certains grands industriels appellerait pourtant de leurs voeux, il s'agit avant tout de protéger nos forêts de prédateurs qui ne voit en elle qu'une opportunité d'exploitation économique soit nécessaire, mais qui ne doit pas se faire, on n'importe quel prix il faudra toutefois réfléchir à ce que l'on pourra proposer à l'avenir aux territoires qui n'ont pas de grands massifs forestiers, mais beaucoup de micro-parcelles qui bien souvent ne font l'objet d'aucun document de gestion de simples associations de propriétaires sont aujourd'hui en train de se créer dans ces territoires et elles font très souvent à ma suggestion avec des structures locales, telles que des PNR ou les pays un excellent travail pédagogique opérationnel de gestion et d'exploitation de ces espaces, elles auront sans doute demain, besoin d'être écoutés sur leur demande. En ce sens au cours des décennies écoulées, la forêt a trop souvent été à bon abordé sous le seul angle du modèle économique ou du Patrimoine familial de nouveaux usages de nouvelles unités sont apparues comme le tourisme, la biodiversité, l'aménagement du territoire, le changement climatique, ceci entraîne inévitablement l'arrivée de nouveaux acteurs qui peuvent eux aussi avoir de nouveaux besoins pour intervenir utilement, ils peuvent avoir besoin de certaines données auxquelles ils n'ont pas accès actuellement, il faudra sans doute dans l'avenir que l'on réfléchisse à la façon de les intégrer un meilleur partage de l'information dès lors qu'il n'y a pas systématiquement une utilisation commerciale de ces informations, mais à ce stade, aujourd'hui, reste 11 ans aux dispositions du présent texte donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et au nom de l'intérêt de la protection de nos forêts constitutif de notre Patrimoine naturel de notre nation, les élus donc du groupe socialiste, écologiste et républicain voteront pour cette proposition de loi. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion, la parole est Marie Évrard pour le groupe RDPI pour 6 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, la forêt a toujours nourri l'imaginaire des rapports de l'homme, la nature selon les sociétés. La forêt occupe une place plus plus ou moins importants dans les représentations sociales des paysages selon que ces derniers soient considérés comme bucolique pittoresque ou romantique, la culture impressionniste de la fin du 19ème siècle là d'ailleurs sublimer la forêt médiéval resurgit et prend une dimension mythique sombre et ténébreuse en double sémantique de l'architecture gothique je pense ainsi à la forêt d'Othe qui s'étend de Joigny dans l'Yonne à Troyes dans l'Aube, sur 28000 hectares et est encadré par des vallées de la vanne de l'Yonne et de l'sont, on l'associe à un pays, le pays d'Othe ce site, je vous invite à le découvrir et composé de sources d'eau à qui l'on accorde des vertus guérisseuse voilà rédemptrice, je pense en particulier aux étangs de Saint-Ange, on note une commune de mon canton. Sur cette représentation enchanté de nos espaces forestiers que nous devons conserver notamment pour s'y promener, mais pas uniquement, outre la beauté de ses paysages si particulier, la forêt, c'est aussi sites à potentiel économique sous-exploité dans ce domaine. Le déficit commercial ne cesse de croître alors même que la France dispose de la 3ème surface forestière d'Europe et de la 1ère place pour ce qui est de la production de Shell cela en partie à cause de la spécialisation de la filière, la forêt est aussi un enjeu environnemental en participant par sa fonction de stockage du carbone à la lutte contre le réchauffement climatique, les surfaces boisées en effet stockent le dioxyde de carbone et rafraîchissent l'air sous l'effet du soleil, l'eau absorbée par les arbres s'évapore, créant de la vapeur d'eau, ainsi des nuages se forment engendrant de nouvelles précipitations et freinant ainsi l'ardeur du soleil mais cette forêt française que nous chérissons tous ces postes potentiel paysager économiques, environnementaux se heurte au morcellement extrêmement de ces parcelles. La grande majorité de la surface forestière française est en effet morcelé entre de nombreux propriétaires privés cette personnalisation à l'extrême de nos forêts et ses conséquences néfastes sur l'environnement, nous l'avons évoqué dans la proposition de loi Jean-Noël Cardoux sous le prisme de l'encrier également à outrance, nous espérons, à ce propos que la navette parlementaire se poursuivra dans un futur proche, plus largement, l'extrême parcellisation du foncier forestier est à la source d'un mauvais entretien des forêts privées d'une sous-sous-valorisation des faux bois et forêts nuisant en définitive à ce que la forêt remplisse pleinement sa vocation environnementale et économique, le texte ici, il ne va pas mettre fin à la parcellisation et ce n'est pas l'objet, à ce titre des Assises de la forêt, dont les conclusions sont attendues prochainement devrait répondre aux défis auxquels elle est confrontée à partir d'une vision partagée de l'ensemble des acteurs de la filière bois, forêts, pour autant, cette proposition de loi pose une Pierre fondatrice pour le renouveau de nos espaces forestiers et en particulier les forêts privées, un certain nombre de ces parcelles appartiennent à des propriétaires qui s'ignorent souvent en raison de leur étage d'un terrain de quelques heures, laisser aujourd'hui à l'abandon, concrètement, beaucoup de ces espaces non entretenues sont inexploitables, tant pour la gestion économique du bois que pour le simple loisir de s'y promener en raison de l'accumulation de Chablis, par exemple l'idée du texte qui nous est proposé de prolonger une expérimentation relatives à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, il s'agit de permettre aux experts forestiers d'accéder aux informations cadastrales numériques relatives aux propriétés forestières, il s'agit d'identifier un ensemble de propriétaires sur un massif forestier et permettre à ses propriétaires de gérer en commun leur sabre de coordonner leur action pour finalement aboutir à une gestion des forêts plus harmonieuse, nous soutiendrons pleinement cette initiative pleine de mon sens et d'espoir pour nos massifs forestiers, beaucoup reste à faire pour notre forêt française une force motrice pour notre environnement et notre économie les constats ont été posées, les solutions sont en train d'être mises en oeuvre, relevons ces défis et en attendant, nous soutiendrons cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Pérenniser une expérimentation revient à reconnaître l'effet positif que le mécanisme apporte dans la vie quotidienne des personnes concernées. C'est une réussite collective que l'on décide d'inscrire dans le long terme. En l'espèce, il s'agit de faciliter le travail des professionnels forestier en leur donnant accès, en leur donnant accès aux données nécessaires à l'exercice de leur mission plus largement le dispositif qui nous est proposée permettra aux acteurs de la forêt française de pouvoir développer une gestion durable de cette forêt. Le groupe, les indépendants et mobilisés depuis plusieurs années sur cette question de la forêt, il a d'ailleurs en novembre 2020, organiser un débat, dans cet hémicycle, intitulé la forêt française face aux défis climatiques, économiques et sociétaux. Les principaux atouts dont nous disposons, grâce à un domaine forestier important importants ont pu être mis en lumière les obstacles auxquels nous devons et devront faire face pour régler les nombreuses problématiques forestières ont aussi été soulevée au 1er rang desquels se trouve le nombre considérable de propriétaires et l'immense diversité des parcelles. C'est précisément ce point qui est traité dans la PPL que nous examinons je souhaite ici saluer nos collègues à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui se sont mobilisés depuis plusieurs années sur ce sujet, ainsi que la rapporteure Anne-Catherine Loisier, dont je connais l'engagement pour les dossiers consacrés à la forêt française et à la filière bois. Les diverses étapes historiques de ce texte ont été rappelés, je ne m'attarderai donc pas à les retracer une nouvelle fois, elles traduisent le travail de conviction des élus pour nos territoires le dispositif prévu par cette proposition de loi, a lui aussi été clairement détaillés précédemment je me bornerai simplement à évoquer 2 sujets majeurs qui me paraissent importants: le 1er concerne l'avis de la CNIL, qui fait partie du processus d'adoption du décret, ce point a été rajoutée à l'Assemblée nationale, le décret en plus de l'application du dispositif traitera de la liste des données qui seront communiquées aux experts forestiers, les données sont toujours un sujet sensible et la CNIL a toute sa place pour faire les recommandations qui s'imposent et effectuer un contrôle. Le second sujet se réfère à l'encadrement très strict et nécessaire du périmètre de l'exception au principe du secret professionnel en matière fiscale que constitue l'accès aux données cadastrales. Ceci étant dit, je ferai un point rapide sur les missions des experts forestiers pour lesquels nous demandons la pérennisation d'expérimentation, en effet, elles ne sont pas des moindres : le travail consiste à la gestion du domaine forestier français, et plus précisément à construire une gestion durable de la forêt. ça suppose évidemment de pouvoir proposer des solutions communes aux multiples propriétés qui dessine un plus grand ensemble et donc de les identifier. C'est aussi et surtout faire cohabiter des considérations environnementales et économiques, fort heureusement, elles ne sont pas qu'on ne peut pas incompatibles, loin de là. Gérer entretenir durablement une forêt, c'est aussi créer une filière bois c'est aussi développé une exploitation intelligente des ressources en bois qui répond aux objectifs français en matière de matériaux cette, enfin, participer à la construction d'une forêt, capable de s'adapter et de lutter contre le dérèglement climatique. C'est pourquoi je partage la nécessité de créer un code de bonne conduite de la filière bois et forêts, le texte présent est le fruit d'un long travail parlementaire de compromis et d'une expérimentation réussie, nous soutenons donc la demande d'adoption conforme qui a été proposé le groupe les indépendants votera en faveur de cette proposition de loi

monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, chers collègues, effectivement, monsieur le ministre, cultiver la forêt cultiver notre forêt, un élément essentiel et ce texte que j'avais eu la chance de rapporter dans la loi ASAP où nous avions déjà eu un accord et je voudrais remercier notre rapporteur Anne-Catherine Loisier du travail qu'elle a réalisé effectivement dans un temps record en termes de en tant que rapporteur mais ce dossier on on on ne peut pas mesurer encore l'impact qui va avoir tellement il est significatif pour nos territoires forestiers, la forêt, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, elle a besoin de femmes et d'hommes sur le terrain, leur donner des moyens à travers ce texte supplémentaire pour être efficaces sur nos territoires, c'est être meilleur sur le renouvellement, que ça soit sur la régénération naturelle, que ça soit sur la replantation ça sera être meilleur sur l'observation, ce que nous avons besoin sur la protection, l'équilibre si voici génétique sur l'aspect sanitaire, Monsieur le Ministre, je souhaiterais qu'on puisse embrasser d'une maire plus volontariste encore sur certains territoires expérimentaux sur la biodiversité et surtout la valorisation combien de propriétaires sont incapables d'aller dire où est leur parcelle forestière combien de surfaces forestières dans tous nos massifs. Sont absolument méconnu de ceux qui en sont les détenteurs et on sait, Monsieur le Ministre, que le gisement de ressources forestières important. Existe dans nos territoires en France et que ce gisement le plus important et souvent Anne-Catherine notre reporter leur le rappel et effectivement se trouve dans la forêt privée se trouvent dans ces parcelles, donc nous avons une capacité, j'ai vécu Anne-Catherine a rappelé. L'époque dans une autre vie, j'étais président de la chambre des lectures, des Vosges, nous avions eu l'audace d'investir dans le cadastre du arriver. Peu de temps avant la tempête, massif des Vosges, le département des Vosges a été celui qui a eu le mois de bois perdus parce qu'on a été capable de retrouver, de démêler tous ces arbres en fonction des différents propriétaires et je dis ça parce que c'est un élément qui est arrivé et qui se reproduira, c'est la vie, et quand on voit les besoins aujourd'hui que nous avons en matière de construction en matière d'ameublement en matière d'isolation en matière de chimie verte embellie en matière de biomasse ce gisement naturel dans nos territoires, qui en plus est un véritable poumon d'oxygène pour nos territoires effectivement ce texte-là qui pourrait sembler comme quelque chose le peu important et absolument significatif parce qu'il vient renforcer tous ces gens et je voudrais dire, Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure des Assises de la forêt, je pense que vous allez bientôt remettre ses conclusions, j'ai eu la chance de de quoi animer d'être présents aux assises régionales du Grand-Est sur la forêt et effectivement c'est une appropriation territoriale et c'est tout le sens de de ce travail, ils étaient présents ces experts forestiers lors de ces assises régionales et parce qu'du fond effectivement et ce sont des acteurs significatifs de l'action forestière au service de des propriétaires, mais de l'intérêt général, aussi, et je voudrais dire à notre rapporteur, que je partage complètement, il serait nécessaire, effectivement, qu'on ait un code de bonnes pratiques cette demande, monsieur le ministre est essentielle pour effectivement qu'on n'assiste pas à la dérive mais qu'on renforce justement au contraire le poids, la présence et le rôle significatif qu'ont ces experts forestiers, dans cette valorisation du poids Thierry Moine de notre Patrimoine. Il y a un autre point, mais on ne va pas l'évoquer, parce que nous souhaitons-le voté conforme, mais c'est sur le sujet que nous avons abordés en commission des affaires économiques, il ne vous faudra évoluer, monsieur le ministre, sur le droit de préférence lorsque vous êtes voisin qui a un propriétaire qui vont, hé bien effectivement, vous êtes prioritaire pour l'acquisition, mais parfois, parce que lorsque vous êtes devenait de plus en plus gros propriétaire vous êtes voisin souvent de partout et ce qui fait que, parfois, de petits propriétaires, voire des communes se trouvent pour priver de leur capacité de faire que cette parcelle, soit un peu plus grande mieux organisés, donne de l'intérêt à ses propriétaires forestiers, donc c'est un autre sujet, mais c'est un sujet sur lequel nous devrons revenir je voudrais tout simplement dire en conclusion, on parle souvent que l'arbre qui cache la forêt, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce texte et qui va être votée, c'est mettre au grand jour, notre forêt et toute son ambition, merci. La parole est à Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité territoire pour 5 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, l'extrême morcellement de la forêt privée, qui représente les 3 quarts de la surface boisée, en France, c'est un frein important et dommageable à une gestion durable de ces forêts et à la mobilisation de la ressource en bois respectueuse des écosystèmes en ce sens l'accès de gestionnaires forestiers aux données du cadastre est un des outils pour améliorer l'information des propriétaires forestiers sur les potentialités de leurs parcelles. Les objectifs de recours accru au bois induit notamment par la réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, la R 20 20 ne seront pas atteints sans la contribution de nombreux propriétaires forestiers, dans le cadre d'une gestion durable, nous aurons cependant une voix quelque peu critique concernant la disposition de ce texte si accéder à une information forestière permettant de gérer en commun des surfaces plus grandes qu'elles ne le sont aujourd'hui, a du sens, la gestion des forêts privées ne doit pas conduire à une gestion exclusivement comptable et à une exploitation intensive à rebours des objectifs climatiques de biodiversité et d'une nécessaire conduite résilientes des forêts face aux menaces sanitaires et au réchauffement climatique. Contrairement à ce qu'indique son intitulé, ce texte permet un accès aux données non seulement aux experts forestiers dont nous ne remettons pas en cause le travail de gestion de la forêt mais aussi aux coopératives forestières qui sont aujourd'hui porteuses souvent d'un modèle d'industrialisation de la gestion de la forêt, nous avons donc là un point d'alerte comme en agriculture, les coopératives ont connu un phénomène de concentration ces dernières années et ont acquis une situation de quasi-monopole pour la gestion de l'exploitation des forêts privées, production de plan et conduite de travaux commercialisation du bois, les coopératives forestières ont intérêt à préconiser aux propriétaires des coupes rases pour mieux vendre ensuite des travaux de plantations sur lesquels se finance, c'est pourquoi nous craignons que l'accès aux données pour ces acteurs favorise une gestion plus industriels de la forêt, monsieur le ministre, vous le savez, la forêt est un et bien plus qu'une simple culture donc nous rejoignons les demandes de la rapporteure sur le code de bonne pratique commun aux 3 familles de gestionnaires concernés ce format ne paraît cependant pas assez contraignant pour pouvoir voter ce texte, nous souhaiterions que l'accès aux données du cadastre soit construite conditionnée à des pratiques sylvicoles réellement durables, notamment via une exclusion des coupera sur de grandes surfaces et de vos plantations mono spécifiques qui ont un effet très néfastes sur la biodiversité sur les sols sur la filtration de l'eau sur les puits de carbone forestier. Les coupera sur de grandes parcelles doivent être doivent être une exception dans la gestion des forêts en cas d'un Pass sanitaire avéré et non une pratique courante il faut encadrer ces procédés de plus en plus contesté par la société civile et les et certains élus locaux, par ailleurs, le petit foncier. Forestiers ne dispose pas de documents de gestion agréés dont les prescriptions pourrait limiter l'intensité des coupes, le nouveau droit accordé par cette proposition de loi devrait ainsi avoir pour contrepartie le respect d'un code de bonne gestion, respectueux de la multifonctionnalité des forêts conçu notamment avec le concours des professionnels, des élus et de l'ingénierie étatique de l'ONF, comme l'avait souligné le député Dominique Potier. En conclusion, il est crucial de respecter la multifonctionnalité de la forêt, la production de bois la forêt loisir, les services écocité écosystémique dont le stockage du carbone, enjeux de ce siècle. La régulation du climat par l'évapotranspiration, la préservation de la biodiversité, malheureusement, aujourd'hui, la forêt et parfois davantage perçu comme un capital dont on souhaite assurer la capacité à fructifier que comme un écosystème vivant à préserver, oui à une gestion responsable durable précautionneuse des forêts, soucieuse des intérêts économiques, mais aussi de la biodiversité, une gestion s'appuyant sur des pratiques de futaie irrégulière et de régénération naturelle quand c'est possible, comptez sur nous pour continuer à défendre un modèle forestier pratiquant une sylviculture douce plus résilientes face au changement climatique mais également plus rentable à terme pour les propriétaires que l'exploitation intensive, dont les travaux sont souvent extrêmement coûteux. Les forêts précèdent les peuples les déserts les suivent, aurait dit Chateaubriand je pense que nous devons chérir nos forêts pourvoyeuse de richesses et d'aménité elle génère l'humus et donc l'humanité est-elle certes disent également d'autres imaginaire donc vraiment la forêt c'est c'est l'essence de nos cultures, donc il faut absolument la préserver et ne pas la cultivé uniquement dans un esprit, un esprit de rentabilité nous conseiller conditionneront donc notre vote aux garantit que le gouvernement pourra nous apporter sur la question des coupes rases et des plantations mono fils spécifique et sur la nécessaire évolution des pratiques forestières, je vous remercie.

C'est le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, un des objectifs de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui est une meilleure connaissance de la propriété forestière privée, objectif que nous partageons en effet les 3 quarts de la forêt française métropolitaine, soit près de 12,6 millions d'hectares appartiennent à 3,5 millions de propriétaires, cela signifie que ce sont des particuliers, des associations ou encore des coopératives qui gèrent eux-mêmes leur forêt mais cela constitue rarement leur activité principale, 60 % d'entre eux possèdent au moins un hectare de bois et n'en tirent aucun revenu, or les parcelles de moins de 25 hectares pour lesquels un plan de gestion n'est pas obligatoire sont globalement peu gérer, voire pas du tout de plus de nombreux propriétaires forestiers, il n'ignore jusqu'à l'existence de certaines de leurs parcelles ainsi l'éloignement géographique des familles et le manque des connaissances sur le milieu forestier conduisit au délaissement de ces petites forêts si ce morcellement contribue à la diversité de la forêt et la protège des dangers l'uniformité, notamment des peuplements espèce l'extrême parcellisation du foncier forestier responsable d'un mauvais entretien de la forêt. Des forêts privées et un frein à une gestion raisonnée des espaces forestiers à la mobilisation du bois, or le propriétaire est un acteur fondamental dans la production de l'espace forestier, la connaissance de la forêt privée passe donc par une meilleure connaissance de ses propriétaires, cette meilleure identification permettrait d'une part une meilleure application du droit de préférence au profit des propriétaires forestiers, voisins en cas de vente d'une petite parcelle boisée, elle permettrait aussi et c'est l'objet de cette proposition de loi, la mise en gestion l'entretien, l'exploitation durable des ressources forestières qui sont caractérisés par un morcellement cela permettrait aussi à développer la production de bois toutefois cette meilleure connaissance et donc cet accès facilité au cadastre pour les gestionnaires forestiers privés doit être soumis non seulement des critères économiques mais aussi à des impératifs de bonne gestion, tels que ceux mis en oeuvre par l'ONF dans le domaine public, c'est pourquoi nous partageons pleinement la nécessité rappelée par le madame la rapporteure de mettre en place un code de bonne conduite, relatif à la protection des données personnelles des propriétaires forestiers et à la protection contre le démarchage commercial abusif, il nous semble aussi important de rappeler que cette action expansion d'accès à certaines données fiscales ne doit pas avoir pour conséquence d'affaiblir la biodiversité, la capacité de régénération des forêts en ce sens, cette connaissance ne doit pas devenir un outil permettant de faciliter les coupes rases et la mal forestation cet accès ne doit pas non plus entraîner la conversion d'un peuplements de feuillus en une plantations mono spécifiques, comme ceux qu'on a pu constater avec la multiplication de la monoculture intensive de sapins de Douglas, un peu partout sur le territoire, en bref, la forêt qui dort ne doit pas devenir une usine à bois dans ce contexte que nous connaissons, où les ressources en bois se raréfie et où les pénuries s'accentue, nous devons y être particulièrement vigilant, on le sait, les arbres sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique et ils ne peuvent déployer leur capacité de stockage de CO2 et de réserves de biodiversité que lorsqu'ils sont en partie intégrante d'une forêt en bonne santé, entretenu malgré ces quelques remarques, nous voterons pour le texte est prolongée cette expérimentation, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est au président Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Merci, Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapport. Faire Anne-Catherine Loisier, mes chers collègues, en tant qu'ancien président de la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen de la loi ASAP je me réjouis de l'examen consensuelle de la présente proposition de loi, en effet, il s'agit, et ça a été dit à plusieurs reprises d'un très bon texte très bon texte sur la forme, il s'agissait de trouver le véhicule législatif adapté à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de cette disposition, considéré comme un cavalier législatif. un texte de bon sens sur le fond, il s'agissait d'une volonté exprimée du législateur de pérenniser une mesure ayant fait l'objet d'une expérimentation à la suite de la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 en effet l'an l'ambition de valoriser nos bois et forêts est largement partagée au sein de cet hémicycle et le Sénat peut se targuer d'être avant-gardiste et force de proposition à la matière, je pense notamment aux travaux du Groupe d'étude présidée par Anne-Catherine Loisier, forêts et filière bois en 2019 ou la commission des finances sur la dite filière en 2015, face à une forêt publique dans l'exploitation est effectivement multifonctionnel, il reste que la forêt privée qui représente, comme vous le savez, 75 % de notre forêt française reste quant à elle, caractérisée par son extrême morcellement qui conduit à sa exploitation aujourd'hui plus de la moitié de la surface forestière privée reste dormante, ce constat n'est évidemment pas un nouveau puisque le rapport mais au B eau de 1978 l'esquissait déjà, et déjà aboutissait à la conclusion que les marges de manoeuvre et de cette filière réside dans la forêt privée mais l'identification des 3,3 millions de propriétaires privés est une difficulté de taille aussi le présent texte en permettant aux experts forestiers agréé d'accéder aux informations cadastrales relève du bon sens, une telle mesure permet de sensibiliser les dits propriétaires et in fine et de mieux répartir l'effort entre forêts privées et forêts publiques la pérennisation de cette mesure, dont l'expérimentation a été concluante permettra, j'en suis sûr un meilleur dialogue entre propriétaires, a-t-elle dialogue est non seulement nécessaire mais également salutaire afin de préserver la multi-fonctionnalité forestière et faire face aux nombreux défis et injonctions diverses que connaît la forêt. Vous me permettrez d'en citer 3 1er défi, le défi économique, celui d'une plus grande adaptation de l'offre de bois de la forêt publique et des forestiers privés à la demande des marchés avec un accroissement de la part des résineux, afin de réduire le déficit commercial de la filière. Le défi écologique bien entendu par le maintien d'un niveau élevé de biodiversité via une importante variété des peuplements de bois mort et d'îlots de vieillissement, l'établissement ou encore la poursuite de pratiques de gestion forestières favorables à la biodiversité. Et le 3ème défi, le défi sanitaire et phytosanitaire, enfin très criant dans mon département, puisque suite à l'épidémie de scolytes et ayant causé le dépérissement de 30000 hectares de peuplement forestier en France, à cet égard est symptomatiquement, je suis convaincu qu'une misère, une meilleure vision d'ensemble, vision d'ensemble public-privé est un meilleur dialogue entre propriétaires de parcelles voisines permet une identification facilité pourrait ralentir la diffusion de scolytes, de surcroît dans un contexte de sécheresse liée au changement climatique lettres et ces raisons, le groupe centriste, soutiendra naturellement cette proposition de loi et je vous en remercie. Merci, cher collègue. La parole est au président Jean-Claude Requier pour 5 minutes pour le groupe RDSE. Président en forme. J'ai le président monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Alors que la France comptait à Miami où ça me drogue d'environ 9 millions d'hectares de surfaces forestières, on estime aujourd'hui que 31 bonsoir la superficie de la métropole est couvert par des forêts, soit 17 millions d'hectares en progression de 0 6 % par à moyenne depuis une trentaine d'années. un goût de % dans ma région, l'Occitanie, cette proportion place notre pays parmi les plus boisé à l'Europe. La forêt française est ainsi à l'évolution constante à l'image aussi il faut le rappeler des modes d'utilisation du bois, en particulier du développement du bois énergie notre foi aujourd'hui au Carrefour de multiples enjeux, des enjeux environnementaux, bien sûr, dans la mesure où les forêts contribuent fortement au stockage du carbone dans le contexte climatique que nous connaissons. juillet de préservation et le développement de la biodiversité, également pour la protection du biotope cabri de nos forêts métropolitaine mais aussi Outre-Mer. Avec une déclinaison gastronomique que j'aimerais situer autour des champignons

sur votre bois dans un contexte mondial de forte spéculation sur les matières premières. Si on a été rappelés près de 3 quarts des forêts appartiennent aujourd'hui à 3 1000000 800000 propriétaires privés, mais la reforestation observée depuis plusieurs décennies, a conduit à morcellement croissant des forêts puisque près de 2 millions de parcelles font moins d'un hectare et presque la moitié des parcelles ne dispose pas d'outils de suivi de la gestion forestière.

l'importance du travail de terrain pour assurer une mise en oeuvre effective du plan de gestion des forêts et les travaux d'entretien de coût pour Yasser Abd ambiance musicale Astral, donc il est question dans la presse un texte au travers du rôle de l'expert forestier et l'indispensable dans en proie à Bienne, donc bien évidemment cette proposition de loi qui vient pérenniser a du positif institué à titre provisoire expérimental par la loi du 13 octobre 2014 puis viendra la main, je veux souligner donc que dans le contexte des Assises de la forêt et du bois en cours. donne la tendance prochainement les conclusions, l'ONF, qui a joué un rôle fondamental de protection du Patrimoine forestier, je tiens à saluer le travail précieux et considérable effectués par l'ensemble de ses agents, là encore l'intervention de la puissance publique a toute légitimité pour aider les propriétaires privés à mieux gérer leurs parcelles au travers l'expertise et de l'information qu'elle peut-il y avoir dit il vous laver avez j'irai plus loin dans la modernisation de notre Patrimoine forestier toutes ses formes, à l'image de ce qu'a pu être le roman agricole, nous ne pouvons plus certes mesuré les limites sur le plan environnemental l'entendement désormais de nouveaux outils, le regroupement des parcelles forestières qui irait plus loin que le droit de préférence les bourses aux échanges nous appelons ainsi de nos voeux, il ne politique ambitieux, il y a pas unification et de gestion forestière, qui irait dans le cadre est plus large d'un développement harmonieux du territoire ruraux dont la forêt n'est qu'une des énormes de ses nombreuses richesses. Merci, cher collègue, la parole est à Serge mais Riou pour le groupe socialiste que le geste républicain pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Puits à carbone espace de loisirs filières économiques la forêt sa gestion, son exploitation sont des enjeux capitaux dans notre pays, trop souvent oubliée des débats la question forestière revêtent une immense importance tant elle constitue une réponse pertinente en nombre de défis que nous devons relever la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à pérenniser une habilitation votée dans la loi d'avenir pour l'agriculture, permettant aux experts forestiers de pouvoir accéder aux données cadastrales pour mener à bien leur mission. Porté par 2 amendements sénatoriaux et mandat émanant des groupes socialistes et centristes cette autorisation d'une durée de 3 ans, leur donner un droit d'accès, sans limitations mais restreint au périmètre géographique d'exercice de leur mission dès 2014 nous avions pressenti la nécessité de faire une exception au principe de secret fiscal pour ces professionnels. Qui concourt notamment à la protection et la mise en valeur des bois et forêts à la préservation de la qualité des sols forestiers ou encore au rôle de puits de carbone des forêts. Le temps nous a donné raison puisque, aujourd'hui, les experts nous demandent le prolongement de ce dispositif en fin de poursuivre leur mission dans de meilleures conditions, cela sera chose faite avec cette proposition de loi qui vient pallier l'échec de l'inscription de cette mesure dans la loi ASAP en 2020. Aussi pourquoi ce prolongement est-il nécessaire, bien qu'elle soit la 4ème forêts d'Europe, la forêt française se caractérise caractérise par son morcellement 12 millions d'hectares de forêts privées 3 1000000 800000 propriétaires avec une moyenne de 3 hectares 40 par propriétaire, le constat est clair dans mon département, la Dordogne, même scénario privé à 98 % la forêt périgourdine est partagé par 90000 propriétaires dans 70000 ne détiennent pas plus de 4 hectares cet émiettement constitue un frein tenace à un usage raisonné et durable des richesses de nos forêts à leur entretien parmi ses nombreux propriétaires et ça a déjà été dit, certains ont parfois même oublié qu'ils en détenaient les dessins à l'abandon, d'autres n'ont pas les moyens nécessaires à l'entretien, ce qui ne permet pas leur valorisation. Pire, la négligence des espaces met en péril notre sécurité en augmentant les risques d'incendie ce manque à gagner à la fois patrimoniale écologique et économique sera je l'espère, en partie, par cette proposition de loi grâce à ce texte, les experts forestiers auront aussi ainsi les moyens pardon d'identifier un un simple de propriétaire sur un même massif forestier pour leur permettre de mettre en place une gestion commune et partagée, les opérations d'entretien et de reboisement seront ainsi facilité, nous pourrons ainsi procéder à une meilleure connaissance et, si nécessaire, rationaliser l'exploitation de notre Patrimoine forestier, je salue le caractère consensuel de ce dispositif, il en va de la pérennité de de la pérennité de nos paysages et de nos modèles agricoles et ruraux, il en va aussi de notre sécurité civile car une forêt mal peu dans un contexte de réchauffement climatique, être sensible au feu et l'envoi de notre résilience économique et de notre capacité de développement, l'importation et la destruction de nos forêts, à des fins d'exploitation sans état d'âme ne sont décidément pas le seul modèle que nous défendons si fièrement merci. Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous le savons, les experts forestiers, les organisations de producteurs gestionnaires forestiers mène des actions d'information à destination de propriétaires sur leurs possibilités de valorisation de leur bois et de leurs forêts, à travers cette volonté autant qu'concourent au reboisement, dans le cadre d'une gestion durable et donc à la fixation et au stockage du dioxyde de carbone, mais vous en conviendrez, pour pouvoir informer ce public, encore faut-il identifier les propriétaires de ces parcelles, ce qu'on appelle pompeusement la matrice cadastrale est le seul instrument qui permet de les identifier, en effet, la forêt française est très morcelée et cette proposition de loi vise à simplifier l'accès des experts forestiers à ces données cadastrales en identifiant les forêts privées, les opérateurs pourraient proposer d'effectuer l'exploitation de parcelles contiguës qui prises individuellement sont souvent trop petites, ce morcellement est un vrai frein à la mobilisation du bois en France et cette loi contribuerait à développer notre production nationale aujourd'hui, les professionnels forestier sont limités par une restriction du nombre de demandes qui peuvent adresser, administration fiscale, c'est la raison pour laquelle une loi de 2014 avait instauré une habilitation temporaire de 3 ans, afin de permettre aux experts forestiers d'accéder sans limitation du nombre de demandes aux informations cadastrales dans le périmètre géographique d'exercice de leur mission. Les experts forestiers ont ainsi pu temporairement bénéficier de cet accès simplifié la fin de sa par ailleurs d'habilitation n'a pas manqué de faire ressurgir l'opacité des propriétés forestières. Le projet de loi ASAP de 2020, chère à notre collègue Daniel Gremillet pour accélération et simplification de l'action publique, entendez résoudre cette problématique en pérennisant cette habilitation par un Arctique adoptée par le Parlement, cependant, ce dernier a été qualifiée de cavalier législatif par le Conseil constitutionnel en décembre 2020 et le dispositif n'a pas été promulguée. Vous l'aurez donc compris la présente proposition de loi entend pérenniser cette habilitation au scènes que législatif dédié L le permis aux experts forestiers aux organisations de producteurs de secteurs forestier et aux gestionnaires forestiers professionnels d'avoir accès sans limitation du nombre de demandes aux données cadastrales dans le périmètre géographique d'exercice de leur mission, ils doivent informer le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes, c'est donner leur sang communiqué afin de leur permettre de mener des actes sur d'information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leur bois et forêts les données recueillies ne peuvent être cédés à des tiers et, enfin, comme l'a dit Madame le rapporteur au décret pris après avis de la CNIL précisera les conditions d'application cette habilitation, ainsi que la liste des données communiquées. Je tiens également à remercier, madame le rapporteur pour la qualité de son travail, je voterai donc ainsi que le groupe, les républicains en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur le ministre. Je souhaite apporter quelques éléments de réponse aux intervenants aux interventions. Oui merci beaucoup monsieur le président, je voudrais simplement compléter mes propos et apporter un élément de réponse à la question de Madame la rapporteure d'abord compléter mais mes propos et notamment mes remerciements que j'ai adressée à Madame la rapporteure également au député Nicolas Turquois qui a porté cette proposition de loi à l'Assemblée,

a eu un véritable soutien transpartisan, ce qui est aussi une preuve de sa totale pertinence deuxièmement apporter un élément de de réponse à Madame la rapporteure et lui dire que je prends ici l'engagement que Metz, équipe a pu la filière dans l'élaboration de ce code de bonne pratique pour lui, l'utilisation des données auxquelles cette loi d'un accès et ses travaux, je crois, vous l'avez dit tout : veiller à la bonne appropriation par des gestionnaires forestiers des des règles fixées dans la loi de décrets d'application et celle rappelée par la CNIL pour l'usage des données, comme vous l'avez dit, dit, et donc répondra ainsi favorablement à votre demande madame la rapporteure. Merci, monsieur le Ministre, la discussion générale est Close, nous passons à discussion du texte de la commission, je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi, le vote sur l'article vaudra vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Monsieur Marc Laménie a souhaité faire une explication de vote. Oui merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, très rapidement, en soulignant tout le travail qui a été fait pour la commission des affaires économiques que l'ensemble des collègues le rapporteur madame Loisier puis aussi félicité déjà la qualité des des interventions vous remercie aussi bien entendu monsieur le. Le ministre mais aussi je étant élus de représentant le département des Ardennes qui fait porte qui est aussi un département forestier, on a quand même aussi, je dirais sur nos territoires, l'attachement l'attachement à la forêt et vous avez évoqué, certes il y a les forêts domaniales, communales syndical et les forêts privées, et c'est vrai que la filière bois le la forêt reste se fait réellement partie du Patrimoine, et je crois que c'est aussi la valorisation du bois et le le morcellement de la propriété, je vois dans le département des Ardennes j'étais maire d'un village suis toujours conseiller municipal, on avait aussi à l'échelle d'un village de 170 habitants sur le morcellement et la la complexité aussi du du cadastre et les difficultés pour je dirais essayer

ce texte a le mérite réellement de trouver aussi des des solutions bon accès des experts forestiers ou de aux données au ou données cadastrales mais c'est aussi sensibiliser et aider aussi beaucoup d'intervenants dans ce domaine en soutenant bien entendu un, comme l'on sur les collègues qui sont intervenus ce texte et on vous remercions. Si cher collègue, je mets donc on voit l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales qui est pour. Qui est contre qui s'abstient m'approprier ce de loi définitivement adoptée, la parole est à monsieur Christian Redon Arazi pour une mise au point au sujet d'un vote. monsieur le président je souhaiterais donc apporter un correctif sur le scrutin, numéro 104 qui a eu lieu le 17 février portant sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives aux compétences de la CEA, donc, monsieur Bernard Jomier ne souhaitait pas voter contre mais voter pour lors du scrutin public numéro 104 je vous remercie donc de bien vouloir enregistrer cette correction. prochaine séance lundi 21 février à 17 heures pour l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française, certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la séance est levée.